occasions de débattre et de légiférer sur notre système de santé ces dernières années. Et pour cause, nous héritons aujourd'hui d'un système de soins dégradé après quarante années de politiques publiques, qui n'ont pas été à la hauteur des enjeux et qui n'ont pas permis d'anticiper les transformations de notre société. La baisse du nombre de médecins engendrée par un beaucoup trop restreint, à des fins de régulation des dépenses de santé, a conduit à la pénurie actuelle. Dans le même temps, le vieillissement de la population, ainsi que l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques ont aggravé la situation.

Je suis surtout convaincue que les tentatives, nombreuses et répétées, de renforcer les obligations des professionnels ne réconcilieront pas les jeunes avec l'exercice de ce métier, devenu peu attrayant, même si dans le contexte actuel, la tentation est grande.

Les agents des trois fonctions publiques, si l'amendement du Gouvernement était adopté, pourraient ainsi réaliser des tâches de secrétariat, gérer l'accueil des patients et effectuer une partie du travail administratif. Pour un jeune qui s'installe, le fait d'avoir à ses côtés, dès le départ, une personne de confiance qui connaît le territoire pourrait avoir un caractère incitatif et l'aider à s'installer rapidement. La rémunération sera versée par l'administration d'origine, puis remboursée par le médecin : il s'agira donc d'une opération neutre pour les finances de la collectivité, en plus d'être facultative et temporaire. Le contrat pourrait également prévoir que le remboursement du salaire soit décalé dans le temps. La commission a souhaité fixer certaines limites, bienvenues, à ce nouvel outil, en créant un dispositif d'amorçage d'une durée maximale de neuf mois, uniquement dans les cabinets libéraux récemment installés, le tout dans le cadre d'une participation du médecin à la permanence des soins ambulatoires. Ces précisions et contreparties devraient rassurer ceux qui craignent de voir les agents publics se substituer durablement aux personnels que le médecin pourrait recruter.

auteurs de ce texte veulent donner des moyens nouveaux et supplémentaires aux élus pour agir en matière de santé, en s'attaquant de manière pragmatique à la question de la charge administrative, qui est un réel problème.

et urbains, étant confrontés aujourd'hui à une démographie médicale en baisse et, donc, à un temps médical devenu très précieux. Face à ce constat alarmant, les élus locaux, de très bonne volonté, se retrouvent bien souvent désemparés. ils continuent d'être force de proposition, afin de créer les conditions nécessaires et favorables à l'installation dans leurs territoires de professionnels de santé et, plus particulièrement, de médecins généralistes. Ce texte s'ajoute à la panoplie des propositions faites au sein de cette assemblée en matière de lutte contre la désertification médicale. d'étendre le dispositif de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux aux cabinets médicaux et aux maisons de santé. Cela permettrait aux médecins souhaitant s'installer dans une zone sous-dotée de ne pas avoir à s'occuper temporairement du recrutement et de la rémunération du personnel administratif.

49 millions d'habitants vivent dans un désert médical, soit 72 % de la population française. Certes, notre population est vieillissante, mais nous avons formé moins de soignants.

Les conséquences de cette politique sont bien connues : allongement des délais pour obtenir un rendez-vous, au risque d'une dégradation de l'état de santé du patient, déport des consultations vers les urgences médicales, difficultés, pour le moins, de trouver un médecin traitant et, donc, rupture du parcours et de la permanence des soins, pourtant garantis par la loi ... Si nous partageons ce constat, nous partageons également la responsabilité de résoudre ce problème. Certaines réponses ont été apportées. Je pense notamment à la création d'une quatrième année d'internat de médecine générale, consacrée à des stages en cabinet médical, en priorité dans les zones médicalement tendues. Cette proposition, formulée initialement par le président Retailleau est de bon aloi et attendue. Toutefois, il nous faut encore en attendre les premiers effets. Mes chers collègues, cette situation nous oblige à accueillir toute initiative avec responsabilité. Il n'est pas question de se priver d'outils qui se révéleront utiles. La proposition de loi examinée aujourd'hui est l'un de ces outils. outils. Déposée par notre collègue Dany Wattebled, elle comporte un article unique qui prévoit la mise à disposition d'agents auprès de cabinets médicaux et de maisons de santé par les collectivités territoriales. En début d'année, lors de ses voeux aux acteurs de la santé, le Président de la République a précisé que « les médecins généralistes doivent pouvoir se concentrer sur la santé, et rien que sur la santé ». Ce texte pourrait permettrait de tendre vers cette ambition. Toutefois, il n'est pas question de déléguer la gestion administrative des cabinets médicaux aux collectivités territoriales. À cet égard, je tiens à saluer le travail du rapporteur, le docteur Daniel Chasseing qui, fort de sa connaissance du monde médical en milieu rural, a su donner à cette proposition de loi une orientation précise. Il faut comprendre ce texte comme l'ouverture d'une possibilité pour les collectivités territoriales volontaristes. Il s'agit de leur donner la faculté de mettre à disposition un agent, pendant une courte période, soit trois mois, renouvelable deux fois, auprès d'un cabinet médical ou d'une maison de santé. Le traitement de l'agent sera naturellement remboursé ultérieurement par la structure d'accueil. Ce dispositif pourrait n'être utilisable que lorsqu'un nouveau médecin arrive, et si celui-ci exerce la mission de service public de permanence des soins. Ce dernier point est très important. La permanence des soins est au fondement de notre réflexion sur la lutte contre la désertification médicale. Elle doit être l'affaire de toutes et de tous. Les élus locaux souhaitent légitimement pouvoir assurer cette mission de service public sur leurs territoires. Nous devons les accompagner dans cette démarche. Vous le savez, mes chers collègues, je suis un ardent défenseur de l'initiative parlementaire. Les expériences sur le terrain, en contact direct avec les élus locaux et nos concitoyens, nous conduisent à élaborer et à proposer des évolutions législatives ayant pour objectif de répondre à des difficultés concrètes. Le texte proposé par notre collègue Dany Wattebled s'inscrit dans cet esprit.

nous leur avons fait confiance quand il s'est agi de mettre en place les agences postales dans une situation similaire ; nous leur avons également fait confiance pour mettre en oeuvre nos décisions lorsqu'il s'est agi de lutter contre la covid-19.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'accès aux soins dans les territoires, particulièrement ruraux, est un problème majeur dont vous avez tous une conscience aiguë- je ne vous apprends rien. Face à cette situation, chaque élu, qu'il soit local ou national, cherche des solutions. Ce sont parfois des propositions de réformes structurelles, parfois simplement des outils pratiques, mais qui peuvent faire la différence et permettre d'accueillir de nouveaux soignants. Dans cet esprit, notre collègue Dany Wattebled, peut-être inspiré par une situation concrète ou par son expérience du terrain, nous fait une proposition intéressante. En prenant exemple sur les partenariats qui ont pu être établis, par exemple entre les collectivités et La Poste, afin de garantir un maillage territorial et une proximité, pourquoi ne pas mettre à disposition d'un cabinet médical ou d'une maison de santé, de façon temporaire et remboursable, un agent communal ? En dépit de leur nombre, les outils financiers et fiscaux, aides de diverses natures déjà en place, ne parviennent plus à déclencher chez les jeunes praticiens la décision d'installation. C'est une vraie difficulté Ces étudiants en fin de cursus, au moment de franchir le grand pas vers l'exercice en autonomie, en indépendance et sous leur propre responsabilité, sont souvent angoissés par des questions pratiques, qui peuvent les amener à reculer. Concrètement, qui pour décrocher le téléphone le premier jour ? Connaître la population locale, le contexte social ? Éventuellement, pouvoir indiquer les lieux et les adresses des patients ? je me souviens, pour avoir accueilli sur ma commune nivernaise un nouveau médecin arrivant de Belgique, de l'aide précieuse de mon adjoint d'alors, facteur retraité, qui l'accompagnait bénévolement dans ses premières tournées.

Lorsqu'un médecin arrive dans une commune, particulièrement rurale, l'équipe municipale au sens large fait un véritable service d'accompagnement dans les premières semaines, et c'est une des conditions d'une installation réussie. Dès lors, permettre la mise à disposition d'un agent public d'accueil connaissant le territoire et ses habitants, afin de faire un lien, aider à la prise de contact pendant une période d'« amorçage », me semble un outil intéressant, et même assez évident. Les soucis d'ordre pratique font partie des critères poussant les candidats à l'installation vers le salariat plutôt que vers l'exercice libéral. Ils nous le disent. Ils apprécient, au moins dans les premiers temps, d'être épaulés et déchargés de certaines contingences matérielles. Évidemment, cette facilité ne réglera pas, malgré son titre prometteur, nos problèmes dramatiques de désertification médicale. Il faudrait pour cela bien d'autres outils, et il faudrait surtout beaucoup plus de médecins, un plan massif de formation. Les médecins sont désormais tellement rares, la pression est devenue telle sur les épaules des étudiants en fin de cursus que ces derniers sont écrasés par les demandes, les attentes, les offres, la responsabilité. On leur propose des primes, des surprimes, des avantages matériels, et dans le même temps on les insécurise, on les terrorise, on les fait fuir. Ce n'est pas en formant 15 % de médecins en plus qu'on sortira de cette surenchère malsaine et contre-productive. Il faut des outils sécurisants, mais surtout une vraie décision politique qui n'a pas encore été prise. Les jeunes Français vont toujours apprendre la médecine en Roumanie ou en Espagne ... Vous aurez compris, mes chers collègues, que cet outil est un outil de plus, et nous y sommes favorables. En l'occurrence, qui peut le plus peut le moins l'expression « maison de santé » sera entendue au sens large, avec ou sans médecin, car il est évident que tous les autres professionnels de santé nous sont également précieux. Infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes, pharmaciens : tous devraient pouvoir bénéficier des mêmes facilités. La parole

La possibilité offerte aux collectivités territoriales de mettre temporairement à disposition un agent public constituerait un nouveau levier d'attractivité médicale pour les territoires, en allégeant les contraintes financières et administratives qui pèsent sur l'installation des médecins.

Malgré les améliorations apportées par le rapporteur Daniel Chasseing pour clarifier le caractère transitoire et temporaire du dispositif, celui-ci appelle des réserves. En effet, le recours aux ressources humaines d'une collectivité locale pour la gestion d'un secrétariat médical soulève de nombreuses interrogations sur la formation professionnelle et les risques d'incompatibilités avec le statut du fonctionnaire, les filières et cadres d'emploi. La proposition de loi ne traite pas la nature des missions qui pourraient être confiées au fonctionnaire territorial. Qu'il s'agisse de la responsabilité juridique de l'employeur et de la garantie du secret médical, le dispositif proposé ne paraît pas d'une opérationnalité optimale. J'ajoute à cela les réserves émises par les associations d'élus locaux lors de leurs auditions sur différents points : les difficultés de recrutement rencontrées par les collectivités dans les métiers susceptibles d'être concernés par la mise à disposition ; le risque de doublon avec d'autres dispositions existantes, notamment la fonction d'assistant médical, ou d'inadéquation entre la formation des personnels mis à disposition et les besoins des cabinets médicaux ; les effets pervers de concurrence entre les collectivités d'attractivité médicale. Outre ces réserves, j'attire aussi votre attention sur les solutions existantes. Je rappelle, par exemple, que nous avons amélioré, simplifié et renforcé la coordination de l'installation des professionnels de santé, en harmonisant les

j'évoquerai rapidement la politique d'attractivité expérimentée en Aveyron depuis 2010 pour inciter les médecins de médecine générale à s'installer. L'implication des médecins en exercice et du Conseil de l'ordre des médecins a été cruciale dans la définition d'une politique d'attractivité médicale qui a emporté, dès ses débuts, l'adhésion de l'ARS. Aborder la désertification médicale recommande une approche globale et partagée à l'échelle d'un territoire. La stratégie repose sur un accompagnement de la profession : d'abord, en favorisant l'accueil de stagiaires par la promotion des terrains de stage, par l'intégration des stagiaires et par une aide financière au transport et au logement des internes éloignés de leur résidence ; ensuite, en soutenant l'établissement de maisons de santé pluriprofessionnelles, adossées à un projet de santé enfin, en créant un guichet unique d'accompagnement à l'installation. Le succès repose sur une coordination inédite de tous les acteurs. La cellule d'accueil des médecins s'est imposée progressivement comme un interlocuteur privilégié. Elle réunit plusieurs acteurs, dans une approche partenariale volontariste et informelle.

de maisons de santé, même si, comme je le dis souvent, le parpaing ne fait, hélas ! pas le médecin ... Ce texte vient donc aider temporairement à l'installation des médecins, en permettant aux maisons de santé et cabinets libéraux

Les médecins manquent partout en France, madame la ministre. Certes, vous n'êtes pas responsable des mauvaises décisions prises par les précédents gouvernements en matière de formation. En En revanche, vous êtes responsable du bon fonctionnement du centre national de gestion- le CNG -, qui, disons-le franchement, ne fonctionne absolument pas ! De par son opacité- aucune information -et son inefficacité dans la gestion des dossiers- les commissions ne se réunissent que très rarement -, le CNG bloque la possibilité pour des milliers de médecins, français ou étrangers, ayant des diplômes hors Union européenne de s'installer dans les territoires, notamment ruraux, s'ils le

Palliez donc le manque d'organisation et de disponibilité des ARS et des jurys du CNG, manque reconnu dans cet hémicycle par votre prédécesseur

Les conséquences sont nombreuses : urgences débordées, renoncement aux soins et, en conséquence, dégradation de l'état médical ou rupture du parcours de soins. Désormais, comme cela a déjà été observé, 72 % de la population habite dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ; 12 % dans un désert médical à proprement parler. Dans mon département de la Haute-Savoie, le phénomène est amplifié du fait de la proximité avec la Suisse, qui entraîne une hausse du coût de la vie décourageant les professionnels de santé à s'y installer, mais aussi une fuite chez nos voisins helvétiques. Certaines communes désespèrent de trouver des médecins. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai remarqué que l'une d'entre elles en était même venue à installer des panneaux à l'entrée du village, indiquant qu'elle cherchait désespérément un médecin généraliste.

ne seront pas tangibles avant quelques années ... Dans l'attente, je suis plutôt favorable à ce que nous prévoyions des dispositifs complémentaires, en particulier s'ils offrent de nouveaux leviers aux collectivités volontaristes sur le sujet. Nombre d'entre elles le sont déjà, malgré le peu d'outils à leur disposition.

Elle ajoute une corde à l'arc des collectivités, et va dans le sens de la décentralisation et de la confiance en nos élus locaux pour être force de proposition. Les modifications adoptées par la commission me semblent bienvenues, car elles viennent border le dispositif dans le but d'en faire une aide temporaire à l'installation de nouveaux médecins, qui pourraient y avoir recours pour un appui administratif ou pour la coordination avec d'autres professionnels de santé du territoire. De même, conditionner la mise à disposition à une participation à la permanence des soins ambulatoires permet de clarifier le lien avec le service public nécessaire à toute mise à disposition. Le fait qu'il s'agisse d'une simple faculté et qu'il n'y ait pas d'impact financier pour la collectivité puisque les salaires devront être remboursés engendre une souplesse qui pourrait être appréciée par les médecins, comme par les collectivités. Par ailleurs, la crainte d'une concurrence entre communes me paraît infondée, dès lors que le dispositif est temporaire et qu'il interviendrait seulement après la prise de décision d'installation

Enfin, avant de conclure, je tiens à insister sur le fait que la mise en place d'outils à destination des collectivités pour participer à la lutte contre les déserts médicaux ne doit pas conduire l'État à se dédouaner de sa responsabilité. C'est à lui que revient en premier lieu le rôle de trouver des solutions, et beaucoup reste encore à faire pour clore ce chapitre. Cela passera nécessairement par une différenciation en fonction des spécificités des territoires, par exemple, pour mon département, la mise en place d'établissements de santé et de formation transfrontaliers, une meilleure prise en charge des soins réalisés dans l'autre pays ou encore une prise en charge des frais de scolarité des personnels de santé en contrepartie d'un engagement à exercer un certain nombre d'années en France. Je suis d'ailleurs, madame la ministre, à votre entière disposition pour échanger sur ces propositions. La parole

sur la désertification médicale, notamment dans les territoires d'outre-mer, où la densité de médecins est très inférieure à la moyenne nationale. Je commencerai mon intervention par une illustration, que ma collègue Victoire Jasmin connaît bien l'année dernière, en Guadeloupe, l'île de la Désirade souffrait d'une absence totale de médecin. Aujourd'hui, malgré l'ouverture récente d'un centre de santé, et la présence quelques jours par semaine d'un médecin, l'offre de soins y demeure très insuffisante et la population rencontre une forte difficulté d'accès

Classée au quatrième rang des régions françaises ayant les densités de médecins généralistes libéraux les plus faibles, la Guadeloupe est donc bien un véritable désert médical. nous misons beaucoup sur les maisons de santé qui se développent dans les communes pour attirer et fidéliser les médecins, et également, dans les prochaines années, sur les premiers résultats de la faculté de médecine de plein exercice aux Antilles. Je tiens à saluer le rapport réalisé par nos collègues Patricia Schillinger et Philippe Mouiller, en octobre 2021, qui préconise de bâtir des centres ou maisons de santé « partenariaux », en étroite concertation entre les élus locaux et les professionnels de santé, ainsi que que le renforcement des liens entre les collectivités territoriales et les facultés de médecine. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, dans le cadre de la niche réservée au groupe Les Indépendants - République en permettant l'élargissement de la liste des entités susceptibles d'accueillir un agent public aux cabinets médicaux et aux maisons de santé. Cette mesure renforcera la boîte à outils mise à la disposition des acteurs locaux pour agir concrètement sur l'accès aux soins. Si nous émettions quelques réserves en commission, nous saluons la réécriture globale de l'article unique sur la proposition du rapporteur, qui permet d'établir un équilibre en encadrant la durée potentielle de recours et en le conditionnant à une installation récente des médecins exerçant en cabinet libéral. Le dispositif a en effet pour principale vocation d'accompagner les médecins à leur arrivée et les inciter à s'installer sur un nouveau territoire. faudra toutefois être vigilants sur les phénomènes de concurrence entre territoires, car il pourrait y avoir un risque que certains d'entre eux multiplient les dispositifs incitatifs, quand d'autres ne pourront rien proposer par manque de moyens. Il ne faudrait pas que la multiplication des dispositifs, sans vision systémique et globale, entraîne une nouvelle hiérarchisation locale. Malgré cela, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera

sa rédaction et son objet pourraient laisser penser, cet amendement ne modifie que très partiellement le dispositif adopté la semaine dernière par la commission des affaires sociales.

des professionnels libéraux et son recours encadré dans le temps. Le seul objet du présent amendement est d'ouvrir la mise à disposition des fonctionnaires auprès de cabinets médicaux ou de maisons de santé en zone sous-dense aux trois versants de la fonction publique, et non plus à la seule fonction publique territoriale. À titre personnel, je n'y voyais que

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Indépendants- République et Territoires. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

vient d'engager l'article 49.3 de la Constitution pour éviter la sanction de l'Assemblée nationale, qui s'apprêtait à rejeter le projet de réforme des retraites. Ainsi, le Gouvernement est seul : les salariés rejettent massivement son texte ; l'opinion publique est vent debout l'unité intersyndicale est totalement contre lui. Et, maintenant, l'Assemblée nationale refuse de s'engager à ses côtés, malgré les tentatives honteuses de débauchage de certains députés. Dans sa solitude, l'exécutif pousse encore plus loin l'autoritarisme. Il a commencé en corsetant les débats avec l'article 47-1. Il finit en interdisant le débat et le vote à l'Assemblée nationale. L'insincérité et l'illégitimité du débat sont totales. Emmanuel Macron et le Gouvernement devront répondre devant le peuple de ce coup de force démocratique. Ce gouvernement ne peut plus rester aux affaires. Il sème le chaos dans le pays. La voix de la raison, la voix de la sagesse, eût été le retrait de ce texte. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE vont renforcer encore leur soutien à toutes celles et à tous ceux qui vont redoubler d'effort dans le pays pour obtenir le retrait de ce projet injuste, ce projet décidé par les marchés financiers. bien ! Acte est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée de la compétence eau et assainissement, présentée par M. Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues

Mes chers collègues, toutes ces initiatives parlementaires relèvent, dans des tonalités et des périmètres différents, bien sûr, l'inadéquation d'un dispositif pensé de manière uniforme, la transformation de la compétence optionnelle eau et assainissement des communautés de communes et d'agglomération en compétence obligatoire. Bon an mal an, ce transfert s'est effectué dans les communautés d'agglomération. dans les communautés de communes, les obstacles s'accumulent. Les conseils municipaux ne cessent de nous alerter par des motions et des délibérations s'opposant à ce qui leur apparaît comme une délégation de compétence beaucoup trop technocratique.

fois, c'est parce qu'aucune solution n'a été trouvée. Il s'agit ni plus ni moins que de la ressource en eau. Devons-nous tourner la tête sous prétexte que les territoires ruraux concernés ne rassemblent pas 76 % de la population ? Ils couvrent, en revanche, la grande majorité des linéaires de cours d'eau à entretenir.

l'assainissement des eaux usées ou à la gestion des eaux pluviales. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement, dite Ferrand, a quant à elle ouvert la possibilité de reporter ce transfert au 1 janvier 2026 pour les communautés de communes. Or, près de cinq ans après ce dernier assouplissement, l'association représentant les intercommunalités de France nous livre un verdict qu'il faut entendre : seul un tiers des communautés de communes concernées exercent à ce jour cette compétence.

», prédisait-il avant de conclure : « Il importait non seulement de laisser ce choix, mais aussi d'apporter une certaine visibilité. » Aurions-nous dit mieux ? Mes chers collègues, devons-nous nous attendre à un mouvement spontané de communes qui opéreraient ce transfert de compétences avant 2026, alors que rien n'a fondamentalement changé ? Je crois assez peu aux propriétés du ruissellement. De même, je ne crois ni aux stratégies d'assèchement financier ni au mariage forcé

concernées ne disposent pas davantage des capacités financières nécessaires pour assumer le plein exercice de cette compétence. Certaines d'entre elles ne souhaitent pas s'engager dans une délégation complexe, avec moult frais cachés qui font ployer la barque.

de la montagne, dite Montagne, qui nous invite à prendre en compte les aménités des territoires montagneux. Ce cadre d'action, c'est la différenciation territoriale. Jacqueline Gourault, alors ministre de la cohésion des territoires, ce principe est garant d'« un État plus agile, plus réactif et plus proche, qui adapte sa réponse et accompagne main dans la main les initiatives des collectivités

C'est vrai : face à une sécheresse structurelle, la réponse ne sera pas uniforme ; elle sera collective. L'Anem, dont je salue le travail, vient de rendre publics les principaux arguments développés par ces maires réticents. Ce sont autant de pistes de différentiation territoriale sur lesquelles il serait- j'en suis sûr -utile de s'appuyer.

Ils relèvent également le risque de doublons, qui implique une forte augmentation des personnels consacrés à ces tâches. Les petites communautés de communes ne pourraient assumer cette charge, si tant est qu'elles réussissent à recruter et à les attirer sur leurs territoires, tant ces métiers sont en tension. Les mêmes élus s'inquiètent surtout des conséquences financières des transferts de compétences prévus : « Les études préalables concluent trop souvent à une forte augmentation du prix de l'eau, difficilement supportable, surtout en période d'inflation.

Or la légitimité des choix politiques en matière de gestion de l'eau passe par une repolitisation de ses instances et le renforcement de l'échelon local de prise de décision. » La gestion différenciée de la compétence eau et assainissement et, au travers d'elle, la bataille contre la sécheresse replacent les élus

de Jean-Yves Roux a une ambition simple. Son article unique vise à supprimer le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes prévu au 1 janvier 2026. Ce texte, qui permet de répondre aux attentes légitimes des élus des territoires ruraux et de montagne, traduit une position défendue de manière constante par le Sénat depuis le vote de la loi NOTRe en août 2015. Vous le savez, en matière d'eau et d'assainissement des eaux usées, le Gouvernement a brutalement remis en cause la liberté des communes par le biais de simples amendements déposés à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi NOTRe. Sénat. Qui a voté la loi NOTRe ? Notre assemblée s'est opposée à ce transfert obligatoire, consciente des difficultés qu'il allait poser aux communes de nos territoires qui ne connaissent pas la même urbanisation que les autres intercommunalités. Toutefois, la commission mixte paritaire (CMP) a trouvé un compromis en reportant le transfert obligatoire au 1 janvier 2020. Par la suite, le Sénat a tenté d'obtenir le rétablissement du caractère facultatif du transfert des compétences eau et assainissement lors de l'examen de différents textes. En effet, dès janvier 2017, le président Retailleau a déposé une proposition de loi visant à rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération. Ce texte a été voté à l'unanimité par le Sénat en octobre 2017, mais les députés ont renvoyé son examen en commission.

Ces différents aménagements n'offrent toutefois qu'un semblant de liberté aux communes, car ils sont limités dans le temps ou dans leurs conditions de mise en oeuvre. Cette situation doit donc évoluer rapidement : l'échéance du 1 janvier 2026 est proche et risque de provoquer un effet cliquet. En outre, les arguments qui justifient la suppression du transfert obligatoire sont toujours d'actualité. On peut notamment évoquer le risque d'augmentation du tarif de l'eau et de l'assainissement, une perte de connaissance des réseaux et une inadaptation du périmètre administratif de l'intercommunalité à la réalité géographique et hydrique des communes concernées.

Au 1 octobre 2022, moins de 30 % des communautés de communes exercent la compétence liée à l'eau et moins de 50 % d'entre elles sont en charge de l'assainissement collectif. Il est évident que les territoires pour lesquels la mutualisation de ces compétences est pertinente l'ont déjà fait depuis plusieurs années, et ce sans attendre que la loi NOTRe le leur impose. Au surplus, l'idée selon laquelle l'intercommunalisation de la compétence eau permettrait de faire diminuer le taux de fuite des réseaux

Les communautés de communes n'obtiendront pas davantage de financements que les communes, de sorte que le transfert de cette compétence n'aura pas d'effet réel sur la diminution de ces fuites. C'est pourquoi l'intention qui anime la proposition de loi de Jean-Yves Roux a emporté la complète adhésion de la commission, qui a néanmoins souhaité améliorer le caractère opérationnel de son dispositif au bénéfice des communes qui souhaitent conserver ou retrouver l'exercice des compétences eau et assainissement. La rédaction qu'elle a retenue entend donc donner son plein effet au principe de différenciation, voté par le Parlement dans la loi 3DS voilà tout juste un an.

faveur. Afin d'éviter aux communes minoritaires de se voir imposer une redescente de compétences qu'elles ne souhaitent pas exercer, il est prévu un mécanisme de transfert à la carte et simplifié des compétences redescendues à la communauté de communes. pour empêcher qu'une minorité de communes se retrouve dans l'impossibilité d'exercer de nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif proposé prévoit que, dès lors lors qu'il existe un accord sur cette demande entre, d'une part, la communauté de communes, d'autre part, une ou plusieurs communes, la restitution peut être opérée. En deuxième lieu, la commission a entendu assurer une stabilité aux conventions de délégation existantes entre les communautés de communes et leurs délégataires. Il ne faut pas remettre en cause des modalités de fonctionnement satisfaisantes pour les communes. Néanmoins, dans l'hypothèse d'un changement du titulaire de l'exercice des compétences eau et assainissement, en raison d'une restitution de ces dernières à la commune, le texte de la commission de la commission permet à la commune de mettre fin à la convention de délégation avant son terme dans le but de la renégocier, d'assurer une restitution effective des compétences aux communes ou de modifier le périmètre des syndicats délégataires. En troisième lieu, la commission a choisi de créer un mécanisme dérogatoire de délégation de compétence plus souple que le droit commun. En effet, les délégataires pourront être des communes ou des syndicats infracommunautaires existants

mesdames, messieurs les sénateurs, votre Haute Assemblée débat aujourd'hui de la question de l'exercice des compétences eau et assainissement au sein du bloc communal. Ce sujet fait l'objet d'un fort intérêt de la part de nos collègues élus locaux. Il est aussi passionnant que passionné et, pour m'être moi-même penchée sur cette question, je sais combien il est sensible dans nos territoires. Et c'est parce qu'il est sensible que le Gouvernement est aussi attaché, depuis dix ans, à ce qu'il soit traité à la hauteur des enjeux qu'il représente.

relève d'une ardente nécessité. Je vais bien entendu, dans le fil de mon propos, justifier cette position. Regardons les choses froidement : quelle est la situation après dix ans d'efforts collectifs tendus vers une meilleure gestion quantitative et qualitative de l'eau ? Aujourd'hui, 14 % des communes appartenant à une communauté de communes exercent encore la compétence eau sans aucune forme de mutualisation.

C'est sur ces 14 % de communes que se portent aujourd'hui toutes nos attentions, soit que celles-ci soient plus durement frappées par les conséquences des épisodes de sécheresse, soit qu'elles estiment ne pas devoir transférer cette compétence à leur (EPCI). Le Sénat s'est déjà saisi de cette question à de nombreuses reprises. Avec le soutien du Gouvernement, il a pu, dans le cadre des lois Engagement et proximité et 3DS, apporter les assouplissements nécessaires pour permettre aux collectivités d'adapter et de différencier les modalités de la gestion de l'eau en fonction des enjeux et des contraintes spécifiques de chaque territoire. Vous estimez que ces assouplissements ne sont pas suffisants et qu'il convient de revenir davantage sur les règles que la loi a fixées voilà plus de dix ans. Si je ne peux que partager, de manière générale et plus encore en l'espèce, votre souhait d'apporter une réponse plus différenciée aux contraintes de chaque territoire, je ne peux non plus passer sous silence ce que la mutualisation nous apporte de façon évidente. : protection de la ressource, sobriété dans son utilisation, qualité de l'eau et meilleure allocation de nos ressources dans la gestion de nos infrastructures.

L'équilibre entre nos prélèvements- 5,5 milliards de mètres cubes par an tous usages confondus -et ce que les cycles de l'eau, petits et grands, restituent aux milieux naturels se dégrade continuellement. Nul besoin de rappeler ici ces faits préoccupants : les épisodes de restriction au niveau de crise sont de plus en plus fréquents : 2 000 collectivités se sont trouvées en tension ou en rupture d'alimentation en eau potable lors de l'été 2022 110 bassins versants, sur le millier que compte la France métropolitaine, sont déjà en déséquilibre quantitatif structurel au mois de février, entraînant des restrictions de consommation dans les territoires concernés. Bref, nous manquons et nous allons manquer d'eau dans les années qui viennent et vous, élus des territoires, êtes sans aucun doute les mieux placés pour savoir ce qu'en seront les conséquences : ... Absolument ! ... c'est le champ que l'on n'irrigue plus, c'est le puits qui manque d'eau, c'est la citerne que l'on doit monter au village. Je sais que vous partagez le constat et l'objectif de protection de la ressource, mais il ne me paraissait pas inutile de commencer par là : s'il y a moins d'eau, il faudra la gérer mieux, et il faudra

garantit pas : nous perdons chaque année 30 % du volume que nous prélevons, ce qui, dans le contexte hydrique que nous connaissons, n'est évidemment pas un facteur facilitant. Actuellement, 170 collectivités ont un réseau dont le rendement est inférieur à 50 %, ce que les techniciens appellent, dans leur jargon, les points noirs de de la gestion quantitative de l'eau. Ce taux de perte est lié à l'état de nos réseaux, lesquels, même si les maires ont fait les meilleurs efforts pour les entretenir, nécessitent encore de lourds investissements. Plus de 40 % de notre réseau devra être renouvelé dans les quarante ans qui viennent. C'est une charge et une dette que nous laissons à ceux qui vont nous succéder, ne nous le cachons pas. Si nous voulons accélérer ces investissements, nous devons le faire ensemble. La sobriété passe aussi par un travail sur les usages : je sais que nos collègues sont, avec les préfets et la profession agricole, très investis pour favoriser une utilisation raisonnable

sans se poser de questions. Or, en 2021, 11 millions de Français ont été alimentés par une eau non conforme. Ce n'est bien sûr pas toujours lié à l'absence de mutualisation, mais l'évidence est tout de même est tout de même que nous assurerons mieux le contrôle de la qualité des eaux en faisant gérer nos ressources par des structures de plus en plus professionnalisées. Le fait est que, dans les services d'eau les plus mutualisés, le taux de conformité microbiologique est excellent. Là encore,

C'est bien selon ce modèle que les maires se préoccupent de leurs réseaux et je veux rendre hommage au travail qu'ils ont souvent fourni, avec les techniciens des eaux, pour assurer l'entretien et la pérennité du réseau. Pour autant, la réalité est là : nous faisons et nous ferons face, dans les trente ans qui viennent, à un mur d'investissements de près de 10 milliards d'euros Toute la bonne volonté de nos élus n'y suffira pas et nous devons trouver les moyens d'investir vite et à la hauteur des besoins. Je me permets de me mettre à la place des maires des 3 600 communes qui n'ont pas encore mutualisé qui doivent donc faire face seuls à ces investissements. Évidemment, ils peuvent avoir accès aux soutiens de la Banque des territoires, donc de l'État, ses agences, mais quelle ingénierie technique et financière ne faut-il pas développer pour souscrire des Aqua Prêts ou remplir un dossier de subvention ! Quelle expertise ne faut-il pas déployer pour poser le diagnostic de l'état du réseau et planifier ses travaux ! Ce n'est pas possible d'entendre cela ! Je fais toute confiance aux maires, mais, soyons lucides, ceux-ci sont et seront plus forts en s'associant à leurs collègues, dans le cadre de l'EPCI, et en mutualisant ressources, moyens et ingénierie.

défi. Ce n'est pas à la loi de le dire ! Vous le savez, le transfert à l'échelle intercommunale vise plusieurs objectifs : redondance et interconnexion des réseaux, mutualisation des moyens humains, techniques et financiers, performance accrue, maîtrise et modernisation des équipements, qualité du service rendu à l'usager.

De ce point de vue, les territoires spécifiques, notamment en montagne, peuvent utiliser les marges et les souplesses prévues par la loi pour adapter la gestion de l'eau à leurs contraintes. Il n'a jamais été question de ne pas le leur permettre. semble, ainsi que l'a d'ailleurs demandé le Comité national de l'eau, que nous avons besoin de donner de la stabilité et de favoriser l'anticipation et la planification. Pour cela, il nous faut nous concentrer, plus que sur la répartition des compétences au sens juridique du terme,

Encore une fois, ne nous leurrons pas : même si de nombreux maires ont géré et gèrent encore l'eau et l'assainissement avec autant de rigueur et de passion, ils ont absolument besoin du collectif pour faire face aux exigences réglementaires, pour mobiliser de l'ingénierie et pour investir massivement dans le renouvellement des réseaux. C'est pourquoi le Gouvernement, investi de la responsabilité de garantir la gestion de la ressource, ne peut revenir davantage en arrière.

de loi de notre collègue Jean-Yves Roux entend rétablir les compétences eau et assainissement dans la liste des compétences facultatives de la communauté de communes. souhaite ainsi revenir sur les acquis de la loi NOTRe, laquelle avait prévu le transfert obligatoire de ces compétences, jusque-là communales à de rares exceptions près, l'échelon de l'intercommunalité. L'ambition du législateur était de maîtriser les coûts et d'offrir aux Français, grâce à la mutualisation des moyens, des services de meilleure qualité. Cette réorganisation territoriale avait suscité à l'époque, et suscite toujours, des inquiétudes chez de nombreux élus, parfois à raison. Trois lois sont venues moduler le dispositif adopté en 2015. Elles ont notamment permis le report de la date butoir de ce transfert au 1 janvier 2026. Vous les avez évoquées à l'instant. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi s'inscrit donc à rebours de ces évolutions. Elle n'est pas pour autant le premier texte présenté au Sénat qui vise cet objectif et, selon toute vraisemblance, elle ne sera Mes chers collègues, nous ne partageons pas cette position, d'abord parce que le transfert des compétences eau et assainissement à l'échelon de l'intercommunalité fonctionne bien.

Nous entendons les difficultés que rencontrent certaines collectivités. Elles sont authentiques et nous ne les contestons pas. Pour autant, la question de la réalité géographique et hydrique, par exemple, qui est souvent citée pour contester cette réforme,

Dans un esprit de stabilité, de continuité, de lisibilité et de clarification des compétences entre les collectivités territoriales, et pour ne pas revenir sur les grands équilibres adoptés en 2015, ... La faute

la question de l'eau est tellement cruciale qu'elle sera sans doute l'un des problèmes politiques les plus complexes et les plus dirimants

survie. Si demain la démonstration était faite que la simple remontée de compétences permettait de régler la question de la pluviométrie dans notre pays, ce qui est tout de même le premier enjeu,

l'occasion de la loi 3DS. La ministre de la cohésion des territoires de l'époque, Mme Jacqueline Gourault, avait pris le temps de nous expliquer le sens de cette différenciation territoriale. Je me permets donc de reprendre ses mots : « Une République différenciée, c'est [ ...] une République davantage décentralisée, où les compétences des collectivités sont confortées et clarifiées. C'est un État plus agile,

Notre rapporteur Alain Marc a travaillé pour améliorer le dispositif proposé. Je salue sa connaissance du sujet et son expertise. Ce texte prévoit de mettre un terme au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement en introduisant

Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Par ces vers empruntés à Boileau, madame la ministre, je veux traduire l'état d'esprit qui nous anime. Vous avez bien compris la détermination, l'opiniâtreté à ne rien lâcher, à ne rien concéder sur ce sujet.

existants, y compris ceux qui sont infracommunautaires, étaient préservés et pouvaient continuer à exercer les compétences. C'est aussi ce que la ministre avait essayé de nous vendre lors de l'examen de la loi 3DS, dont j'étais corapporteur avec Françoise Gatel. Or à y regarder de plus près- c'est subtil

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour évoquer ensemble le sujet, récurrent dans notre hémicycle, du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Je tiens tout d'abord à saluer, cher Jean-Yves Roux, votre initiative d'inscrire ce sujet ô combien important à notre ordre du jour. Celle-ci s'ajoute aux initiatives de nos collègues Mathieu Darnaud et Jean-Michel Arnaud. À la réticence des élus locaux et du Parlement, différents motifs censés justifier la nécessité de ce transfert ont été opposés. À titre d'exemple, je citerai l'urgence de réduire la dispersion des compétences ou encore l'importance d'abaisser le taux de fuite des réseaux.

en ce qu'il ne coïncide pas du tout avec la réalité hydrique et géographique du terrain. Comme l'a rappelé notre rapporteur Alain Marc, dont je salue le travail, ce passage de flambeau engendre une perte de compétences à l'échelon local, mais aussi une hausse des dépenses publiques locales du fait du recrutement de nouveaux agents dédiés. La commune reste dans certaines situations l'échelon le plus satisfaisant pour exercer les compétences eau et assainissement. À plusieurs reprises, le Parlement a tenté de revenir sur le caractère impératif de ce transfert.

C'est tout particulièrement le cas dans les territoires les plus ruraux et de montagne. D'après une publication récente d'Intercommunalités de France, seulement 48 % des intercommunalités exerçaient la compétence eau en octobre dernier. Ce chiffre illustre bien les difficultés ressenties sur le terrain pour faire face à ce transfert imposé au forceps. Plutôt qu'une approche uniformisée, nous souhaitons privilégier une réponse sur mesure adaptée aux besoins et aux spécificités des territoires. Il convient de faire confiance aux élus locaux. Le texte amendé par la commission et notre rapporteur apporte la souplesse nécessaire et permet de répondre à tous les cas de figure qui se présentent à nous. En permettant un transfert à la carte des compétences eau et assainissement, cette proposition de loi donne aux communes la marge de manoeuvre indispensable pour mener sereinement leur mission

Adopter cette proposition de loi, c'est faire confiance aux maires. Adopter cette proposition de loi, c'est faire vivre les principes de différenciation et de subsidiarité en s'appuyant sur une dynamique de liberté locale. Le groupe Les Indépendants - République

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons aujourd'hui vise à faire figurer de nouveau les compétences eau et assainissement dans la liste des compétences facultatives des communautés de communes.

Par respect du principe de subsidiarité, nous jugeons légitime que des élus puissent librement choisir de mettre en commun, ou non, les compétences eau et assainissement et décider des modalités de cette mise en commun selon les particularités de leur territoire. En matière de gestion de l'eau, les questions relatives à la géographie et aux capacités techniques se posent nécessairement. Souvent, le périmètre administratif de l'intercommunalité ne se superpose pas à la réalité hydrique du territoire. Je pense notamment aux territoires ruraux et aux territoires de montagne,

Car oui, la multiplication des épisodes de chaleur et de sécheresse nécessitera de plus en plus de mises en commun pour éviter les conflits d'usage autour de l'eau. À ce titre, je souhaite revenir sur la question centrale

sous-investissement gonflent et gonfleront les prix de l'eau au détriment des usagers. Aujourd'hui, 1 million de foyers sont déjà concernés par une facture d'eau d'un montant supérieur à 3 % de leurs revenus. Si l'on peut soutenir l'intelligence des élus territoriaux et respecter leur faculté de faire les meilleurs choix pour leur commune, on peut aussi souligner la nécessité de mutualiser et d'investir collectivement. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires se partagera sur ce texte entre quelques votes pour et une majorité d'abstentions, mes collègues estimant que cette proposition de loi n'est pas la réponse aux problèmes évoqués.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans la vie législative- nous ne le savons que trop -, de simples amendements peuvent avoir une immense portée. C'est en effet par un simple amendement gouvernemental au funeste projet de loi NOTRe, en 2015, sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État, que le gouvernement d'alors avait fait adopter le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux EPCI, y compris dans les communautés de communes. Face à l'opposition farouche de l'Association des maires de France et d'une bonne partie du Sénat, nous avons depuis obtenu de haute lutte un certain nombre d'assouplissements : plusieurs reports de la date de transfert, finalement fixée au plus tard au 1 janvier 2026 sous conditions, la possibilité de déléguer la compétence à un syndicat ou à une commune par la loi du 3 août 2018 et la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019.

Nonobstant ces différentes mesures d'adaptation législative, le résultat final ne semble pas avoir répondu totalement aux inquiétudes des élus de la ruralité et de la montagne, car il ne résout pas le problème de fond la loi oblige toujours les communes à transférer l'eau et l'assainissement à leur communauté de communes. La mise en place de cette communautarisation généralisée a été voulue, nous dit-on,

La loi NOTRe se donnait ainsi pour objectif une mutualisation efficace des moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, notamment dans les zones rurales. Nous y voilà, les mots magiques sont lâchés : « rationalisation, maîtrise, mutualisation, circulez ! » Combien d'inepties génératrices de gabegie d'argent public ont été inventées sur la base de ce mirage ? Comment un principe aussi général peut-il être opérant au vu de la très grande hétérogénéité des situations locales ? L'Assemblée des communautés de France de France (AdCF) a constaté que, à la fin de 2021, seules 33 % des communes avaient effectivement transféré aux communautés de communes la compétence en question. À l'évidence, la fixation du niveau d'exercice de cette compétence ne peut être uniforme et déconnectée du terrain, mais doit relever de considérations matérielles et techniques propres à chaque territoire. Cela vaut encore davantage pour les territoires ruraux, où les modalités de gestion d'un service public peuvent varier d'une commune à l'autre et nécessiter de maintenir une gestion directe par la commune ou les syndicats en place afin de permettre une capacité d'intervention plus souple et plus efficace. Que dire encore des investissements coûteux et des recrutements qui seraient nécessaires à la seule mise en oeuvre de ces transferts, si tant est qu'ils ne soient pas contestés par la Cour des comptes, sans réel bénéfice en termes d'efficacité pour les territoires concernés ? À n'en pas douter, ces transferts s'accompagneraient dans certains cas d'une hausse importante du prix de l'eau qui concerne les communautés de communes, les auteurs de la présente proposition de loi entendent privilégier une approche pragmatique, moins coûteuse et technocratique, adaptée aux réalités géographiques et hydrologiques des territoires. Suivant l'essence même du principe de subsidiarité, il reviendrait aux communes de décider du niveau d'exercice de ladite compétence en matière d'eau et d'assainissement. Nous sommes donc impatients de connaître la position du Gouvernement et, par la suite, l'avis de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement finira-t-il par accepter de revenir sur une disposition profondément contestée sur le terrain ? Le fait qu'à peine un tiers des communautés de communes se soient vu transférer la compétence eau, presque dix ans après la loi NOTRe, montre que les maires restent prudents sur le sujet, ce qui devrait suffire à faire réfléchir le Gouvernement. Pour conclure, et avant même d'examiner le texte proposé par nos collègues du groupe RDSE, que je remercie, il me semble indispensable de préciser un point technique qui peut prêter à confusion lorsque l'on évoque, sans autre précision, l'eau et l'assainissement. Le réseau d'eau potable est sous pression et peut donc avoir n'importe quel périmètre. En revanche, les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sont gravitaires. L'eau potable est facturée, comme l'assainissement des eaux usées, une redevance pour la collecte, le transport et l'épuration. Au contraire,

Les élus locaux ne veulent pas, à juste titre, que la compétence eau et assainissement soit gérée à l'échelon intercommunal. Les conseils municipaux souhaitent conserver ce levier, qui a aussi une dimension sociale.

que des contraintes géographiques. En effet, la qualité et la quantité de ressources disponibles tout comme l'éloignement du lieu de captage, qui génère une certaine longueur de canalisations, et les conséquences liées à la nature des sols sur le vieillissement des canalisations ont un effet sur les coûts de production et d'entretien. Il faut aussi prendre en compte le fait que, dans les zones rurales, l'habitat dispersé oblige à se doter d'un réseau de distribution de grande longueur. Les coûts d'entretien par habitant des réseaux de distribution et de collecte ne sont pas les mêmes qu'en agglomération. Comment une intercommunalité pourrait-elle gérer de façon efficiente ce type de difficultés ? Vous comprenez bien que la réponse du Gouvernement, par votre voix, madame la ministre, le 24 janvier dernier, pour défendre le principe du transfert sans l'ombre d'un argument fondé, comme vous venez de le faire, ne me convient pas. Mais je ne pense pas que vous soyez responsable de cette situation. Je crois plutôt que c'est encore une conséquence négative de la fameuse loi NOTRe.

cette compétence obligatoire. De plus, ce transfert nécessitera la création d'un service au sein d'une communauté de communes,

nous entretenons nos réseaux et tout se passe bien en qualité et en volume. C'est une petite commune industrielle, dont de nombreux habitants ont des salaires modestes ; nous sommes heureux et fiers d'offrir l'eau à un coût très bas, bien en dessous de la moyenne, autour de 1 euro.

Il faut, à l'image de ce que le Gouvernement veut promouvoir, notamment la décentralisation et la différenciation, que l'on puisse tenir compte des réalités des territoires : la mutualisation

de la commune à une communauté d'agglomération. Avant ce transfert, le pétitionnaire déposait en mairie son permis de construire, laquelle envoyait la demande d'avis au syndicat intercommunal d'eau potable, qui renvoyait son avis à la commune une semaine après. Aujourd'hui, avec le transfert à la

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

sur cette base que certaines d'entre elles ont été créées ou assemblées voilà quelques années. Je ne connais pas un élu, madame la ministre, pas un maire qui se désintéresse de la gestion de l'eau dans sa commune. Pas un ! C'est probablement la compétence la plus importante exercée par nos élus locaux. Ils ont développé une connaissance de ces réseaux à nulle

Loin de justifier leur opposition au transfert obligatoire par le seul désir de conserver à l'échelon communal une compétence supplémentaire, les élus locaux avancent des arguments de fond. Ainsi, ils insistent sur l'importance de conserver une gestion de proximité des réseaux et d'assainissement dans les territoires où l'habitat est dispersé et où la densité de population au kilomètre carré est faible. Au quotidien, l'entretien des réseaux est assuré par les agents techniques, mais aussi, souvent, par des élus bénévoles, comme cela a été dit. Élus et techniciens ont acquis une connaissance des réseaux et une réactivité qui permettent d'assurer un service de qualité à un faible coût pour les usagers. Le transfert de la compétence à l'intercommunalité suscite des interrogations sur la capacité des agents de la communauté de communes à assurer les travaux de surveillance et d'entretien, ainsi que la gestion des pannes, sachant qu'il faut souvent plus d'une heure en temps normal pour se rendre au siège de la communauté de communes et que les déplacements sont très difficiles, parfois impossibles, en hiver. Les usagers devront également se déplacer ou toutes les questions. À long terme, la perte d'expertise des techniciens et des élus communaux et l'absence de transmission de cette expertise conduiront à dégrader encore plus le service aux usagers. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des études préalables et des témoignages recueillis une augmentation des prix de l'eau, liée notamment à l'harmonisation des prix à l'échelon intercommunal et au surcoût en équipements et en masse salariale qu'entraîne une gestion intercommunale. Les conséquences financières du transfert de la compétence ne sont pas négligeables. Ces études concluent à une forte augmentation des prix de l'eau difficilement supportable, surtout en période d'inflation, pour les ménages à faible revenu et pour les agriculteurs montagnards, très dépendants de l'eau et déjà économiquement fragilisés. Les élus de montagne s'inquiètent aussi de la gouvernance dans la gestion des compétences eau et assainissement dans les intercommunalités où les communes de montagne ne sont pas majoritaires et où les spécificités de leurs problématiques ne sont pas prises en compte ni même parfois comprises. Madame la ministre,

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, présentée par M. Bernard Fialaire et plusieurs de ses collègues

les dernières années ont été marquées par la révélation de nombreuses affaires de faux. Si le phénomène des fraudes artistiques n'est pas nouveau, il semble aujourd'hui en pleine expansion. La hausse de la demande, l'explosion des prix sur le marché de l'art et l'essor de la vente d'art en ligne contribuent sans doute très largement à doper et à faciliter ce type d'escroqueries. Aucune forme d'art n'est épargnée et la nature des fraudes se diversifie. Loin de se réduire à la fabrication de fausses oeuvres d'art, ces fraudes prennent aussi la forme de faux certificats attestant d'une fausse authenticité, mais aussi, de plus en plus, d'une fausse provenance.

Il est donc important que nous disposions d'outils efficaces pour prévenir et réprimer ce type d'infractions. Le problème, c'est que le seul texte de nature législative dont nous disposons en France pour réprimer spécifiquement les fraudes artistiques est un texte daté, d'application limitée et aux effets peu dissuasifs. Il s'agit de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, plus connue sous le nom de loi Bardoux. Son champ d'application ne correspond plus à la diversité des oeuvres d'art que l'on trouve aujourd'hui sur le marché et, par conséquent, à la diversité des faux. Il concerne uniquement les catégories d'oeuvres d'art en vogue à la Belle Époque- peinture, sculpture, dessin, gravure, musique -et laisse de côté les faux manuscrits, fausses photographies, faux meubles ou faux objets de design, ainsi que les oeuvres d'art que les oeuvres d'art numériques, qui soulèvent de nombreuses difficultés en matière de respect des droits de la propriété intellectuelle. Au sein de ces catégories déjà très limitées, la loi Bardoux ne vise que les faux qui correspondent à des oeuvres authentiques qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Elle n'est donc pas applicable aux faux qui concernent des oeuvres anciennes, en dépit du nombre important d'affaires en la matière. Enfin, le texte en vigueur ne s'intéresse qu'aux faux revêtus d'une signature apocryphe. Il exclut donc tous les faux sans signature, à l'instar des faux « à la manière de », ainsi que tous les faux sans auteur identifié, dont relèvent pourtant l'essentiel des arts premiers, des antiquités, de l'art médiéval, de l'art islamique, des arts asiatiques ou des arts appliqués. À cela s'ajoute le fait que les peines prévues par la loi Bardoux ne sont pas assez sévères pour être dissuasives. Elles sont de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Il n'est en outre pas possible de les alourdir, quelle que soit la circonstance dans laquelle l'infraction est commise. Il y a bien un autre texte spécifique aux fraudes artistiques : le décret Marcus, datant de 1981, qui vise à réprimer les tromperies sur l'authenticité d'une oeuvre d'art et d'un objet de collection. Néanmoins, ce texte ne s'applique qu'aux transactions : il permet de sanctionner les seuls vendeurs contrevenants d'une amende d'un montant maximal de 1 500 euros. Il est vrai que plusieurs infractions de droit commun peuvent être utilisées pour poursuivre les auteurs de fraudes artistiques. Je pense en particulier aux délits de contrefaçon, d'escroquerie, de tromperie ou de faux et usage de faux, qui sont beaucoup plus lourdement sanctionnés. Mais, comme aucun de ces délits n'est propre au marché de l'art, leur champ d'application n'est pas parfaitement adapté pour assurer la répression des fraudes artistiques dans leur globalité. La caractérisation des faits se révèle complexe pour certaines natures de faux ou dans certaines circonstances, notamment lorsque le faux n'a pas fait l'objet d'une quelconque transaction. C'est pour combler les insuffisances du cadre juridique en vigueur que j'ai déposé, en décembre dernier, avec mes collègues du groupe RDSE, la proposition de loi dont nous débattons ce soir portant réforme de la loi Bardoux. Nous nous sommes appuyés sur les différentes réflexions conduites sur le sujet au cours des dernières années. La Cour de cassation a notamment consacré un colloque à ce sujet en 2017 l'Institut Art et Droit, une association de réflexion réunissant juristes et acteurs du monde de l'art, a mis en place un groupe de travail à compter de 2018. Le résultat de ses travaux a été présenté lors d'un colloque en mars 2022 et a inspiré notre proposition de loi. Notre texte propose la création d'une nouvelle infraction pénale dans le code du patrimoine, destinée à remplacer celle qui est prévue par la loi Bardoux. Afin de mieux appréhender la diversité des phénomènes de fraudes artistiques, nous avons décidé de faire porter la matérialité de l'infraction non plus non plus sur le nom ou la personnalité de l'artiste, comme le prévoit la loi Bardoux, mais sur les atteintes portées aux oeuvres d'art elles-mêmes, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent et que l'auteur de l'oeuvre authentique soit ou non identifié ou identifiable. C'est la raison pour laquelle le texte, tel qu'il a été déposé, prévoit de sanctionner la réalisation, la présentation, la diffusion ou la transmission, à titre gratuit ou onéreux, de tout bien artistique ou objet de collection qui serait, par quelque moyen que ce soit, affecté d'une altération de la vérité sur l'identité de son créateur, sa provenance, sa datation, son état ou toute autre caractéristique essentielle, et ce sous réserve qu'elle ait été faite en pleine connaissance de cause. Afin d'améliorer la prévention et la répression des fraudes artistiques, nous avons veillé à durcir suffisamment l'échelle des peines. À titre principal, nous avons proposé d'aligner celles-ci sur celles qui sont applicables en matière d'escroquerie, de recel ou de blanchiment, soit cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Nous avons proposé qu'elles puissent être alourdies à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ou lorsqu'il est commis de manière habituelle. Nous avons prévu enfin qu'elles passent à dix ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. À titre de peine complémentaire, notre texte autorise la confiscation du bien ou de l'objet saisi ou sa remise au plaignant. Elle rend également possible cette confiscation ou cette remise en cas de relaxe ou de non-lieu, lorsqu'il est établi, à l'issue de la procédure judiciaire, que le bien ou l'objet saisi est affecté d'une altération de la vérité. Ces dispositions ne changent pas le droit existant. Comme la création de cette nouvelle infraction rend obsolètes les dispositions de la loi Bardoux, l'article 2 l'abroge et opère les coordinations afférentes dans le code général de la propriété des personnes publiques, seul texte de valeur législative au sein duquel cette loi est mentionnée. Maintenant que je vous ai exposé les raisons qui nous ont amenés à déposer cette proposition de loi, permettez-moi de vous présenter la position de la commission de la culture sur ce La proposition de loi lui paraît répondre à une véritable attente, exprimée aussi bien par les artistes ou leurs ayants droit, que par les professionnels du marché de l'art, les praticiens du droit et les services enquêteurs. Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Claude Marin, n'avait-il pas lui-même appelé, en 2017, à repenser intégralement le délit même de fraude artistique ? Ces fraudes ne portent pas seulement atteinte à des intérêts privés, ceux des acquéreurs lésés, ceux des artistes dont les droits sont bafoués, elles érodent également la confiance dans le marché de l'art et les institutions patrimoniales et constituent, finalement, une menace pour la création. La commission est donc convaincue qu'une réforme de la loi Bardoux est indispensable afin d'améliorer la protection des acquéreurs et le respect des droits des artistes, de restaurer la crédibilité du marché de l'art et d'accroître la transparence et la fiabilité dans ce secteur. Le fait que la proposition de loi prévoie de réprimer les atteintes portées aux oeuvres d'art elles-mêmes plutôt que de chercher à réparer le seul préjudice subi par les acquéreurs ou les auteurs des oeuvres authentiques, comme dans la loi Bardoux, présente à ses yeux un double avantage. D'une part, elle permet de ne plus conditionner l'infraction ni à la nécessaire identification d'un artiste ni à celle d'une transaction ou d'un cadre contractuel ; d'autre part, elle revêt un caractère hautement symbolique en ce qu'elle est une manière d'affirmer que les oeuvres d'art ne sont pas assimilables à de simples marchandises, mais qu'elles constituent, au contraire, un bien commun à tous. La création d'une infraction spécifique aux différents types de fraudes artistiques envoie un signal fort aux auteurs de ces fraudes sur le caractère hautement répréhensible de leurs actions. La proposition de loi permet de corriger les principales lacunes de la loi Bardoux. Elle élargit le périmètre de l'infraction aux falsifications affectant l'ensemble des oeuvres d'art, quel que soit leur support, sans la restreindre à certaines catégories d'oeuvres particulières ni distinguer entre les oeuvres selon qu'elles sont encore ou non couvertes par les droits patrimoniaux de l'auteur authentique. Elle étend l'infraction aux falsifications relatives à la datation, l'état ou la provenance d'une oeuvre d'art, sans la limiter aux seules falsifications liées à la signature ou à la personnalité de l'artiste. Elle alourdit considérablement le régime des peines et rend possible leur aggravation dans certaines circonstances, tout en restant dans une échelle comparable à ce qui est prévu en matière d'escroquerie, de recel ou de blanchiment. Ce niveau apparaît cohérent compte tenu de l'implication croissante des réseaux criminels en matière de trafic d'oeuvres d'art. La commission a aussi souhaité clarifier la rédaction de certains aspects de la proposition de loi pour garantir son caractère pleinement opérationnel. Les auditions ont en effet mis en évidence un certain nombre d'ambiguïtés de la rédaction initiale, incompatibles avec l'exigence de précision imposée par la matière pénale ou susceptibles de nuire à la qualification des faits. Je pense ainsi à l'emploi de la notion de « bien artistique », jugé trop risqué dans la mesure où aucun code ni texte ne la définit ni ne l'utilise. Je pense aussi à la notion d'« altération de la vérité » employée dans le cadre du délit de faux et usage de faux, qui pourrait se révéler inopérante en matière artistique tant la vérité est souvent difficile à établir en ce domaine, comme en témoignent les fréquentes querelles entre experts. Notre objectif n'est ni d'empêcher à l'avenir les experts d'émettre une opinion ni d'entraver la liberté de création des artistes en rendant impossible la pratique de la copie, du plagiat, de la parodie ou du détournement d'oeuvre d'art d'art dès lors qu'il n'y a pas d'intention de tromper autrui en faisant passer l'oeuvre ainsi créée pour ce qu'elle n'est pas. La commission a décidé de recentrer l'infraction sur les différents types de comportements frauduleux destinés à tromper autrui sur et autour de l'oeuvre d'art. La définition de l'infraction a été totalement revue et distingue désormais quatre hypothèses. La première hypothèse est celle de la réalisation ou de la modification d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection dans l'intention de tromper autrui sur l'identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition. Cette définition reprend les éléments rendus obligatoires par le décret Marcus sur les certificats d'authenticité délivrés par les vendeurs à l'occasion des transactions. Elle permet de sanctionner l'auteur ou le commanditaire du faux proprement dit. La deuxième hypothèse est celle de la présentation, de la diffusion ou de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d'un faux en toute connaissance de son caractère trompeur et sans rétablir la vérité à son sujet. Elle vise à sanctionner le receleur. La troisième hypothèse est celle de la présentation, de la diffusion ou de la transmission d'une oeuvre ou d'un objet authentique en mentant sur l'identité de son auteur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition dans l'intention de tromper autrui. Elle vise à sanctionner l'escroquerie sur l'authenticité de l'oeuvre, même en l'absence de remise de fonds. La dernière hypothèse est celle de la présentation, de la diffusion ou de la transmission d'une oeuvre ou d'un objet en lui inventant une fausse provenance. Elle vise à sanctionner l'escroquerie sur la provenance de l'oeuvre ou de l'objet, peu importe que celui-ci soit authentique ou faux. La commission s'est également attachée à clarifier la rédaction des dispositions destinées à permettre au juge de mettre hors circuit les oeuvres et objets qui seraient reconnus comme des faux. Les auditions ont révélé à quel point cette mise hors circuit constitue une question complexe. À la fois, il est à n'en pas douter essentiel que les faux artistiques soient détruits ou retirés par quelque moyen que ce soit pour éviter qu'ils ne reviennent tôt ou tard sur le marché, mais, en même temps, force est de reconnaître que la question du faux n'est pas totalement binaire : comment être certain qu'une oeuvre constitue un faux, en dehors des faux grossiers, par exemple ceux qui ont manifestement été réalisés après la mort de l'artiste qui en serait prétendument l'auteur ? ? Peut-on considérer qu'une oeuvre d'atelier signée de la main du maître est un faux ? Est-il possible de porter atteinte au droit de propriété, garanti par la Constitution, en confisquant une oeuvre lorsque celle-ci appartient à un propriétaire de bonne foi ? question qui a conduit en 2021 la Cour de cassation, dans une affaire dite Chagall, à confirmer la décision de la cour d'appel qui avait ordonné l'apposition de la mention « Reproduction » sur une oeuvre contrefaisante avant sa restitution à un propriétaire, plutôt que de demander sa destruction. Cette décision suscite l'incompréhension des représentants des artistes au regard des atteintes aux droits privatifs de l'auteur. Elle illustre bien toute la difficulté de cette question. question. La commission a donc souhaité mettre à la disposition du juge un panel d'outils pour écarter définitivement les faux des circuits commerciaux : la confiscation de l'oeuvre ou de l'objet, sa destruction ou sa remise à l'artiste victime de la fraude ou à ses ayants droit. Sur ma proposition, la commission a choisi de ne pas faire mention du marquage, de peur que le juge ne retienne systématiquement cette option qui, pour être moins attentatoire au droit de propriété, n'apporte aucune garantie réelle d'un retrait définitif de l'oeuvre ou de l'objet du marché. la commission n'a pas souhaité imposer au juge le retrait systématique des oeuvres du marché. Il ne s'agit que d'options à sa disposition. La rédaction retenue lui laisse la possibilité, en fonction des circonstances d'espèce, d'ordonner l'une ou l'autre de ces solutions, ou de n'en rien faire, parce que toutes les oeuvres ou objets litigieux ne sont pas nécessairement des faux intégraux. Certains peuvent revenir sur le marché dès lors que leurs véritables caractéristiques sont rétablies. Pour compléter ce dispositif, la commission a décidé de mettre en place un registre des fraudes artistiques, sur lequel auraient vocation à être inscrits tous les faux reconnus comme tels qui ne seraient pas détruits.

Pour finir, la commission a très largement complété le dispositif de la proposition de loi en matière de sanctions. Elle a prévu les peines applicables en cas de commission des faits par une personne morale. Elle a élargi le champ des circonstances aggravantes, pour répondre à l'émotion suscitée par plusieurs affaires récentes, comme celle des faux meubles de Versailles, qui a d'autant plus choqué l'opinion que son auteur était un professionnel extrêmement reconnu et qu'il a fait du tort à l'une de nos plus prestigieuses institutions patrimoniales. Il nous a donc semblé justifié d'alourdir également les peines applicables lorsque les faits portent préjudice à un établissement public relevant de l'État ou d'une collectivité territoriale ou lorsqu'ils sont commis par des professionnels du marché de l'art. par cohérence avec l'introduction de cette seconde circonstance aggravante, nous avons également autorisé le juge à prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercice à titre temporaire ou définitif de l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle, ou à l'occasion de laquelle, l'infraction a été commise. Il s'agit d'une peine complémentaire fréquemment prévue pour ce type de délits : on la retrouve, par exemple, en matière de tromperie. L'ensemble des améliorations apportées par la commission au texte initial avait pour but de garantir une meilleure répression des fraudes artistiques, dans le souci évident d'en améliorer aussi la prévention. Nous espérons que la suite de la discussion parlementaire permettra encore d'enrichir ce texte. Nous attendons beaucoup des conclusions de la mission sur les faux artistiques conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui devraient être rendues en juillet prochain. Nous avons largement échangé avec le président du Conseil supérieur, ainsi qu'avec les responsables de cette mission. Nous savons qu'une partie de leur réflexion porte sur les différentes procédures judiciaires qui pourraient être mises en place pour lutter contre la prolifération des faux sur le marché. Ils envisagent notamment d'ouvrir une voie d'action civile, complémentaire à l'action pénale que nous proposons. Cela existe en matière de contrefaçon. Je pense, par exemple, à la procédure jugée très efficace de saisie-contrefaçon. Ils voudraient également proposer des solutions afin de mieux encadrer l'activité des plateformes en ligne. Nous considérons que ces pistes pourraient donner un intérêt supplémentaire à la présente proposition de loi, en offrant des possibilités complémentaires d'action à l'encontre des faux. besoin de moyens d'actions judiciaires rapides pour intervenir contre les pratiques frauduleuses de certaines galeries éphémères ou de plateformes en ligne se fait de plus en plus sentir. Au-delà de la réforme de la loi Bardoux, il nous paraît indispensable de mieux sensibiliser les services de la police et de la justice aux spécificités des infractions qui peuvent être commises dans le domaine de l'art et de renforcer les moyens mis à la disposition de ces services pour que la lutte contre les fraudes artistiques gagne en efficacité.

Cette proposition de loi permet d'aborder un défi majeur pour l'ensemble du secteur du marché de l'art : la lutte contre les faux artistiques. Qu'est-ce qu'un faux artistique ? Vous l'avez dit, au sens large, il s'agit d'un objet destiné à passer pour autre chose que ce qu'il est réellement. réellement. Le but est de tromper l'acheteur en faisant passer cet objet pour une oeuvre authentique. Si ces fraudes ne constituent pas un phénomène nouveau, on constate ces dernières années une multiplication sans précédent des transactions illicites et l'apparition de nouvelles formes de falsifications d'oeuvres d'art, notamment liées au développement des plateformes en ligne. Je souhaite saluer le travail mené par l'Office l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, compétent pour diligenter les enquêtes, y compris les plus complexes, et celui de la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), qui contribue pleinement à la réflexion et à la sensibilisation sur ce sujet si important. Les faux artistiques constituent en effet un véritable fléau, qui porte atteinte aux intérêts des professionnels du marché de l'art, mais aussi et surtout à ceux des acheteurs, des auteurs et de leurs ayants droit.

Si plusieurs autres infractions de droit commun, comme la contrefaçon, l'escroquerie, le faux et usage de faux, permettent également de sanctionner les coupables de telles fraudes, ce texte apparaît aujourd'hui daté, car il présente des lacunes et n'est plus adapté au marché actuel Ces lacunes sont de plusieurs ordres. La liste des oeuvres falsifiables est réduite aux seules oeuvres de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique. Elle ne permet pas d'appréhender la diversité des oeuvres d'art d'aujourd'hui. Je pense à la photographie, aux arts appliqués, mais également à l'ensemble des nouvelles formes d'art numérique, dont les frontières ne cessent d'être repoussées, comme le montre le développement NFT l'incrimination de fraude artistique est limitée aux seules oeuvres « non tombées dans le domaine public », alors même que les oeuvres anciennes suscitent une part très importante des affaires de faux. Enfin, les sanctions prévues par la loi Bardoux- deux ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende -peuvent sembler peu dissuasives. Je partage donc l'avis du rapporteur : oui, la loi Bardoux mérite d'être actualisée. Le ministère de la culture en est pleinement conscient et le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), placé sous l'égide de mon ministère, s'est emparé de ce sujet l'an dernier, l'an dernier, confiant à MM. Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, deux éminents spécialistes, une mission visant à évaluer l'opportunité d'une évolution du cadre juridique actuel pour mieux définir le faux en art, faciliter sa détection et renforcer sa répression. Les résultats de cette mission seront connus définitivement en juillet prochain. Le présent texte propose plusieurs évolutions de la loi pour répondre à cette forte attente d'actualisation et la rendre plus opérationnelle. Il prévoit notamment l'élargissement du périmètre de l'infraction aux falsifications affectant l'ensemble des biens artistiques et objets de collection, afin de protéger l'ensemble des supports l'alourdissement des peines, afin de les aligner sur celles applicables en matière d'escroquerie ; ou encore l'extension de l'infraction aux falsifications relatives à la datation, l'état ou la provenance d'une oeuvre d'art, pour ne pas la limiter plus aux seules falsifications liées à la signature ou à la personnalité de l'artiste. Plusieurs évolutions ont été apportées lors de l'examen du texte en commission la semaine dernière, afin de prendre en compte les échanges et remarques formulées au cours des auditions. Ces dispositions vont dans le bon sens. Nous sommes pleinement convaincus de la nécessité de faire évoluer cette loi pour renforcer la lutte contre la fraude en matière artistique.

La directive européenne d'avril 2022 interdit de cumuler deux dispositifs dérogatoires différents. Dès lors, quelles sont les possibilités ? Si nous voulons maintenir un taux de TVA sur la seule marge à la revente,

un taux de 20 % sur la marge. Des expertises et simulations sont encore nécessaires pour avancer vers cette possibilité. C'est pourquoi, avec Gabriel Attal, nous venons de lancer une concertation avec les professionnels du secteur, pour qu'une décision soit prise avant l'été. L'objectif est d'aboutir à une disposition qui sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2024, afin qu'elle soit examinée par le Parlement cet automne, ce qui permettra d'achever, d'ici à la fin de l'année 2023, la transposition de cette directive. Soyez en tous cas assurés que la ministre de la culture que je suis, comme l'ensemble du Gouvernement, suit très attentivement ce dossier et demeure très attachée à la compétitivité et au dynamisme du marché de l'art français, qui représente 50 % du marché de l'art de l'Union européenne ! Vu le nombre de galeries internationales qui s'installent à Paris, le dynamisme de nos musées, le succès des foires et la vitalité de la scène de l'art contemporain de notre pays, la France est véritablement aujourd'hui au centre du marché européen. Elle doit le rester. Elle peut le rester. La parole

Mais là où l'histoire devient mordante, c'est qu'il n'agit pas ainsi dans le but de s'enrichir : il donne, gratuitement, ses faux aux musées qui, pendant plus de vingt ans, ne remarquent rien. Finalement démasqué par un conservateur perspicace, il fera l'objet d'un documentaire,, diffusé en 2015 au cinéma. Et, quand il est interrogé sur la tromperie à grande échelle qu'il a orchestrée, il a cette sentence déconcertante : « Je n'ai commis aucun crime ! comprendre par là qu'il n'a pas bénéficié d'un enrichissement personnel. Cette histoire romanesque témoigne de l'acuité de la présente proposition de loi et de la nécessité de mieux appréhender, culturellement et juridiquement, le faux en art. Car ce qui apparaît principal dans la défense de Mark A. Landis, en l'occurrence l'absence d'enrichissement personnel, n'est en réalité que secondaire ; ce qui est central, c'est la vaste duperie qui a abouti à ce que des institutions culturelles présentent au public pendant des années de fausses oeuvres d'art. En France, la loi Bardoux, accompagnée du décret Marcus du 3 mars 1981, semble désormais dépassée, obsolète pour traiter efficacement du faux. Il est évident qu'à la Belle Époque, et même il y a quarante ans, le faux en art ne revêtait pas les mêmes formes qu'aujourd'hui, devenues plus sophistiquées et plus étendues.

il est indispensable d'actualiser la loi pour mieux lutter contre les fraudes artistiques. Mais par-delà la modernisation de notre arsenal législatif, la philosophie même de la proposition de loi est extrêmement contemporaine. Celle-ci ne se contente pas de viser les auteurs de l'infraction et la réparation des préjudices subis, elle tend surtout à protéger les oeuvres d'art en tant que telles. Autrement dit, l'oeuvre d'art, et la prévention des atteintes qui pourraient lui être portées, devient l'objet même de la C'est un renversement de paradigme très intéressant et radicalement moderne dans son approche. Ainsi, de nombreux questionnements se posent, de plus en plus, autour de l'oeuvre et de sa vie. C'est particulièrement vrai dans la filière musicale, où l'une des conséquences du numérique- qui n'était pas la plus attendue -a été de redonner un élan, voire même parfois une existence, à des oeuvres qui semblaient condamnées à l'oubli. En d'autres termes, il n'y a plus de parcours uniforme, linéaire pour une oeuvre ; et, plus encore qu'auparavant, la vie d'une oeuvre se trouve décorrélée de celle de son auteur- ce qui rend sa protection d'autant plus impérieuse. D'autre part, le postulat de cette proposition de loi est aussi une déclinaison de l'exception culturelle, tant soutenue par la France : une oeuvre d'art n'est aucunement un bien et, à ce titre, elle doit disposer de protections spécifiques. C'est précisément ce raisonnement qui avait conduit la France et d'autres pays européens à créer un droit d'asile des oeuvres en 2015 et 2016, lorsque les destructions et pillages d'oeuvres et de monuments parfois plurimillénaires se multipliaient dans les territoires sous domination de l'État islamique. Nous avions alors été nombreux, y compris sur ses travées, à nous émouvoir et nous révolter contre ce qui constituait un effacement méthodique de sociétés, de cultures, d'histoires, de croyances, d'imaginaires, en somme de vies et de faits qui sont constitutifs d'une certaine vérité historique et anthropologique. La question de la vérité a été au coeur de nos riches échanges sur ce texte. S'il est aisé de s'accorder sur le principe que le faux est éminemment une altération de la vérité, il est beaucoup plus délicat d'apprécier cette altération en matière artistique.

Mais de plus, l'état des connaissances et des techniques nous oblige à l'humilité, notamment devant le développement des oeuvres créées par l'intelligence artificielle. Des expériences ont déjà prouvé qu'avec le degré de technicité actuel les conservateurs et spécialistes de l'art peuvent se retrouver démunis pour distinguer une oeuvre authentique et un faux façonné par une machine informatique. Plutôt que de nous en remettre à la notion instable d'altération de la vérité, nous avons préféré caractériser précisément le faux et l'infraction qui s'y rattache, élargissant à cette occasion son spectre par rapport à la loi Bardoux, afin de renforcer l'effectivité et la portée du dispositif. Enfin, j'aimerais évoquer une préoccupation majeure : la confiance. L'implication la plus dangereuse et déstabilisante du feuilleton Landis, et de tout faux qui circule de manière générale, c'est la défiance qui en résulte, aussi bien sur le marché de l'art que dans le rapport aux institutions culturelles. Quoi qu'il en soit, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi constitue un premier pas important pour moderniser notre corpus législatif. Nous devrons impérativement rester très vigilants face aux développements de l'art numérique, où les défauts de preuve d'authenticité et les risques de falsification sont, par définition, accrus. À n'en pas douter, comme dans beaucoup de secteurs, le numérique et

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il fallait une certaine intrépidité pour partir à l'assaut du vénérable édifice constitué par la loi Bardoux. Les premiers coups de pioche donnés, vous vous aperçûtes que ses fondations, encore bien solides, pouvaient expliquer la durabilité d'élévations que l'on pensait croulantes. Avec l'humilité qui vous caractérise, vous reconnaissez que la proposition de loi que vous nous soumettez est encore imparfaite. Elle a néanmoins le mérite de définir le cadre utile d'un chantier de reconstruction. Il restera à M. le sénateur Agénor Bardoux bien d'autres mérites- dont celui d'avoir participé à la révision du texte de. La loi de 1895 intéresse le droit des contrats. Dans le domaine particulier du marché de l'art, elle apporte des garanties à l'acheteur en le préservant du dol, de l'escroquerie et de la falsification. Son objet n'est pas de protéger l'auteur ni son oeuvre, mais de sanctionner les tromperies sur l'authenticité d'une oeuvre pour donner à l'acquéreur une assurance de délivrance conforme. Elle met en oeuvre pour cela deux notions essentielles, l'intentionnalité de la fraude et l'authenticité de l'oeuvre. À l'usage, ces deux principes sont parfois apparus d'établissement complexe la question de l'authenticité recoupe souvent celle de la provenance et l'intentionnalité est quelquefois difficile à établir quand elle est l'enjeu de controverses académiques. Le décret modifié du 3 mars 1981, dit décret décret Marcus, a tenté de corriger ce défaut en introduisant des gradations dans le degré de certitude de l'authentification. Les formules qu'il propose - « attribué de l'école de », du « style » ...- ont eu le mérite d'offrir au vendeur la possibilité de ne pas engager totalement sa responsabilité quand il estimait que l'authenticité pouvait être discutable. Néanmoins, de nombreuses questions restaient pendantes, comme celle relative à la révision de la valeur d'une oeuvre à la suite d'une nouvelle attribution. que la Cour de cassation, par son deuxième arrêt Poussin, a considéré qu'elle n'était pas créatrice de qualités nouvelles, mais révélatrice de qualités préexistantes, ce qui permettait au vendeur de dénoncer le contrat. Par ailleurs, la loi Bardoux était inspirée par une conception très académique des beaux-arts, qui fut rapidement dépassée par l'évolution de la pratique artistique. En 1913, Marcel Duchamp expose sa roue de bicyclette et, plus tard, sa fontaine, en posant la question : « Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas d'art ? ». En l'occurrence, ce qu'interroge Marcel Duchamp, c'est le statut de l'artiste et de l'oeuvre, et c'est dans ce questionnement que réside la démarche artistique. La notion d'authenticité n'a alors plus aucun sens. Avec cet exemple est rapidement abordé le problème juridique complexe des relations entre la législation du patrimoine et celle de la propriété intellectuelle. L'auteur conserve des droits sur l'oeuvre même après sa vente. Comment établir l'authenticité d'une oeuvre que son auteur aurait reniée et qu'il aurait peut-être détruite ? Monsieur le rapporteur, à plusieurs reprises dans cet hémicycle, notamment lors de la discussion sur les lois de restitution, vous avez exprimé vos interrogations d'ordre philosophique sur la valeur de la notion de propriété appliquée à une oeuvre d'art. Dans l'exposé des motifs de votre proposition de loi, vous considérez que l'oeuvre appartient d'abord à une culture avant d'appartenir à un individu. L'abrogation de la loi Bardoux est alors pour vous un moyen de nous inciter à une réflexion plus profonde.

Une oeuvre d'art authentique. Une oeuvre de dentelle, ou d'orfèvrerie juridique, pour filer la métaphore. Car elle nous entraîne dans un univers de droit où chaque concept doit être bien pesé et où la subtilité le dispute à la finesse. Monsieur Fialaire, en tant qu'auteur et rapporteur de ce texte, vous me permettrez de vous dire : chapeau l'artiste Votre proposition réforme la loi Bardoux, du nom de l'honorable sénateur inamovible Agénor Bardoux, aïeul d'une personnalité chère à la famille politique dont je suis membre, à savoir l'ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing. En proposant ce texte en 1895, Agénor Bardoux avait réagi au scandale provoqué par une escroquerie artistique dont avait été victime Alexandre Dumas fils. Ce dernier avait acquis un tableau qui lui avait été vendu comme étant un Corot et qui était en réalité une oeuvre de Paul Désiré Trouillebert trente ans plus tard, les arnaques artistiques font toujours la une des gazettes : faux sièges de Marie-Antoinette acquis par le château de Versailles, fausse Vénus de Cranach achetée par le prince de Liechtenstein et, surtout, acquisition par le Louvre Abu Dhabi d'une stèle de Toutankhamon illégalement sortie d'Égypte en 2011. Trois exemples qui montrent à quel point la fraude artistique est non seulement d'actualité, mais même en plein boom. Trois exemples qui montrent aussi à quel point elle peut être protéiforme. Frauder, ce n'est pas seulement mentir sur l'authenticité d'une oeuvre. Cela peut tout aussi bien être mentir sur son origine. Et cela peut concerner des objets de toute nature et de toute époque. C'est cette extension du domaine de la fraude que ne couvre pas la loi Bardoux. Depuis 1895, la création artistique a changé, tout comme le marché de l'art et l'art des escrocs. Ce texte ne protégeait que les oeuvres d'art classiques, telles que les peintures ou les sculptures, mais pas les photographies, les objets de design, et encore moins la vidéo et les NFT. De plus, elle ne protège que les oeuvres les plus récentes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. La loi Bardoux était dépassée depuis longtemps. À l'heure de la numérisation de l'art et de son commerce, sa survivance a presque quelque chose de poétique. Mais poésie ne rime pas toujours avec effectivité juridique ... Le principal apport du texte qui nous est proposé est d'élargir la répression de la fraude à la réalité contemporaine du phénomène, phénomène, à l'ensemble des oeuvres aujourd'hui concernées, signées ou non, contemporaines ou anciennes. L'arsenal juridique dont nous disposons à côté de la loi Bardoux ne permet-il pas déjà de remédier à ses lacunes ? C'est là que l'on entre dans le byzantinisme. Le code pénal sanctionne bien les délits de contrefaçon, d'escroquerie, de tromperie et de faux et usage de faux. Mais le pénal n'est pas le civil. De même, le décret Marcus de 1981 de 1981 ne permet de sanctionner que les vendeurs contrevenants. Les trous dans la raquette sont donc importants. L'autre grand apport du texte est de revaloriser la peine encourue. La loi Bardoux n'est pas assez sévère : deux ans et 75 000 euros d'amende, sans modulation en fonction des circonstances, compte tenu de l'ampleur des trafics actuels, c'est très insuffisant. Nous ne pouvons que soutenir le renforcement substantiel de ces sanctions, qui sont alignées sur les infractions d'escroquerie, recel ou blanchiment. Cela portera la peine et l'amende à cinq ans et 350 000 euros pour les cas ordinaires et permettra de monter à dix ans de prison et 1 million d'euros d'amende quand les faits sont commis en bande organisée.

De plus, les apports du CSPLA, qui semble travailler sur les procédures judiciaires qui permettraient de mieux lutter contre les faux sur le marché de l'art, seront sans doute parfaitement complémentaires avec le travail effectué sur la présente proposition de loi.

Non seulement on ne peut jamais être sûrs qu'un faux en est bien un, mais, de plus, un faux peut être beau, un faux peut être une vraie oeuvre d'art. Face à cet épineux problème, monsieur le rapporteur, vous avez refusé la solution grossière de la destruction systématique. C'est sage ! Vous avez aussi refusé celle du marquage, au motif qu'un marquage peut toujours être escamoté. Vous proposez donc la mise en place d'un registre des faux artistiques. C'est la solution qui nous semble la plus pertinente. Mais, parallèlement, vous déléguez au juge le soin d'apprécier ce qu'il devrait advenir du faux en fonction des circonstances de l'espèce. Comme trop souvent, le législateur se dessaisit. Ne peut-on au moins utiliser notre compétence pour énumérer de manière restrictive les conditions dans lesquelles un faux devrait être détruit ou confisqué ?

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, dite loi

De ces génies d'autrefois aux délinquants de notre temps, il n'en demeure pas moins qu'à l'ancienneté de la réponse du droit doit être opposée la modernité des pratiques des faussaires. C'est en cela que résident l'enjeu et l'objectif de la proposition de loi présentée par Bernard Fialaire et cosignée par les treize autres sénateurs du groupe du Je rappelle que ce texte désuet, à l'application limitée, aux effets peu dissuasifs, inadapté aux enjeux contemporains du marché de l'art international, cristallise la frustration des ayants droit et professionnels du marché de l'art.

Le monde de l'art a ses propres usages, ses propres traditions, et il n'est pas évident de se positionner de façon tranchée entre ce que le droit peut accepter et ce qu'il doit interdire. La liberté de la création est essentielle à l'art. Elle est ce que la liberté d'expression est à la pensée. Cet équilibre fragile entre la nécessité de protéger les oeuvres contre leur exploitation frauduleuse et le principe intangible de liberté de création doit donc être recherché en priorité.

Le faux artistique ne devrait-il pas être pensé comme une atteinte à la vérité- et de surcroît à l'intérêt général -plutôt que comme une atteinte à un intérêt particulier ?

Nous souhaitons ainsi affirmer que les oeuvres d'art ne sont pas assimilables à de simples marchandises, mais qu'elles constituent un bien commun. Ce bien commun pourrait s'étendre demain non plus aux seules catégories d'oeuvres d'art et d'objets de collection en vogue à la Belle Époque, mais à toutes les nouvelles formes de création, d'aujourd'hui et du futur. et du futur. La fraude serait désormais étendue aux falsifications relatives à la datation, à l'état ou à la provenance de l'oeuvre d'art et ne serait plus limitée aux seules falsifications liées à la signature ou à la personnalité de l'artiste. Si la finalité est d'améliorer la protection des consommateurs, de restaurer la crédibilité du marché de l'art et d'accroître la transparence et la fiabilité dans ce domaine, reste la difficulté inhérente à l'art d'appréciation de l'altération de sa vérité, tant la vérité en matière artistique est souvent difficile à établir et sujette aux aléas des connaissances et des techniques. Je finirai en soulignant le signal fort que cette proposition de loi adresse aux auteurs de fraudes artistiques sur le caractère hautement répréhensible de leurs actions. Si la loi Bardoux se distingue par ses effets peu dissuasifs, l'alourdissement du régime des peines devrait contribuer à rendre toute sa crédibilité à notre marché de l'art- qui occupe le quatrième rang mondial -et à protéger les amateurs d'art contre la tromperie, tout en garantissant la liberté de création des artistes. Le groupe du RDSE se félicite par ailleurs des modifications et enrichissements apportés par la commission. Il votera bien évidemment cette proposition de loi.

alors qu'en réalité il avait été peint par un artiste bien moins renommé de l'école de Barbizon, Paul-Désiré Trouillebert. Ce scandale a abouti à la loi Bardoux, qui, depuis sa promulgation en 1895, n'a jamais été modifiée et continue d'être appliquée par les juges. Toutefois, on constate ces dernières années une multiplication des fraudes en matière artistique, ainsi qu'une augmentation considérable des transactions illicites. Face à ces dernières, cette proposition de loi pointe à juste titre les insuffisances des dispositions juridiques

est trop restrictif pour couvrir toute l'étendue des faux dans leur réalité actuelle. Elle ne vise en effet que les arts existant à la Belle Époque tels que la peinture, la sculpture, le dessin, la gravure ou la musique, alors que de nouvelles formes artistiques- photographie,

obsolète, enfin, car l'échelle des peines n'est plus en adéquation avec les infractions similaires, comme les délits de contrefaçon ou de faux et d'usage de faux. Comme le souligne justement la proposition de loi, le recours aux dispositifs existants, comme ceux qui

les auteurs et leurs ayants droit, les acheteurs- amateurs d'art ou investisseurs -, les professionnels du marché de l'art, ainsi que les institutions dont l'activité se trouve parasitée, sont ainsi dans l'attente d'une réforme.

On peut déplorer à cette occasion que la lutte contre les faux en matière artistique n'ait pas été jusqu'alors une priorité, en comparaison des efforts engagés à l'égard des contrefaçons dans d'autres secteurs économiques. Bernard Fialaire s'est attaché

À partir des travaux menés en commission, plusieurs amendements ont été adoptés en vue de clarifier les nouvelles règles et d'éviter certains effets collatéraux relevés lors des auditions. L'approche retenue place au centre du dispositif non plus les droits qui lui sont attachés, mais l'oeuvre en elle-même. entre protection des oeuvres et liberté de création. La définition de la fraude artistique a été réécrite en ce sens, afin de ne pas entraver les usages non frauduleux de l'oeuvre d'art. Pour lutter contre la multiplication des fraudes, la commission a aussi prévu l'alourdissement des peines en cas de circonstances aggravantes, lorsque la fraude est commise par un professionnel du marché de l'art ou lorsque le préjudice est subi par une collectivité publique. Le juge pourra par ailleurs prononcer une interdiction d'exercice de l'activité professionnelle ayant conduit à l'infraction. La question du sort de l'oeuvre falsifiée est également traitée par le texte issu des travaux de la commission, qui s'en remet au juge pour décider la confiscation, la restitution ou la destruction de l'oeuvre.

Certes, nous sommes conscients qu'une loi ne suffira pas à résoudre tous les problèmes posés par l'évolution du marché de l'art, notamment celui de la circulation des oeuvres l'activité des plateformes en ligne si peu réglementée. Ce texte constitue néanmoins la première pierre de ce chantier et adressera un signal fort aux auteurs de fraudes artistiques.

est encore aujourd'hui le texte de référence en matière de fraude artistique. Pourtant, avec l'évolution des escroqueries et la diversification des pratiques artistiques, elle est devenue lacunaire. Le droit en vigueur n'apporte pas de réponse satisfaisante face à la prolifération des cas de fraude artistique, dont témoigne l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. La loi Bardoux limite l'incrimination à certains types de cas. Premièrement, elle ne concerne que les oeuvres de peinture, sculpture, dessin, gravure et musique. Cette considération énumérative de l'art est aujourd'hui très limitée au regard de la grande diversité de la création artistique. l'oeuvre d'art en question doit présenter une signature apocryphe ou un nom usurpé. Or les pratiques de falsification sont de plus en plus complexes et imaginatives. Troisièmement, enfin, l'oeuvre ne doit pas être tombée dans le domaine public, ce qui relègue dans l'oubli un vaste pan de l'art. Les peines prévues par la loi de 1895 en cas d'infraction sont bien trop faibles et éloignées de celles qui sont prévues par d'autres dispositifs similaires, visant par exemple à réprimer la contrefaçon. Il est donc nécessaire de muscler l'arsenal de réponse à la fraude. Notre pays représente le second marché de l'art dans le monde. Cela nous engage à veiller avec exigence à la transparence et à la fiabilité des acteurs. Il nous faut rétablir la confiance en nos institutions culturelles, nos artistes, nos experts, nos lieux de vente, meurtris ces dernières années par de nombreux cas d'escroquerie. Rappelons la tristement célèbre affaire des faux meubles achetés par le Château de Versailles entre 2008 et 2012 à plusieurs professionnels du marché de l'art, pour un montant total de 2,7 millions d'euros. Une réforme de la loi Bardoux, texte précurseur, mais aujourd'hui daté, se révèle donc nécessaire, afin de protéger au mieux le marché de l'art français et ses institutions, tout en rassurant les acquéreurs et les artistes.

qui ont mis en lumière le caractère éminemment complexe de la réponse à apporter aux évolutions des fraudes artistiques. Se pose notamment la question de la protection des créations artistiques numériques,

Ce texte va dans le bon sens. Par son adoption, le Sénat donnera le coup d'envoi d'une vaste réflexion sur la prise en considération des évolutions de l'art et du droit d'auteur. sera également nourrie au mois de juillet prochain par les conclusions de la mission lancée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Ses apports permettront notamment de mieux définir le faux en art et de simplifier sa détection,

Paul-Désiré Trouillebert, lui, est toujours vivant. Peut-être lit-il alors, dans les colonnes des journaux, les conclusions du débat parlementaire, dont l'une de ses toiles fut à l'origine, parce qu'elle avait été attribuée à un autre, à savoir à Corot.

De l'amertume, à ne devenir pour l'histoire qu'un copiste de Corot ? Du cynisme, à observer le comportement moutonnier du marché de l'art, transformant les artistes en brevets et plaçant, surtout, au second plan l'émotion esthétique produite par la contemplation d'une toile

qui ne prévoit pas de réhabilitation pour l'auteur véritable de l'oeuvre. Vieille de plus de cent ans, cette loi nécessitait une actualisation pour adapter les moyens de la lutte contre les faux artistiques aux nouvelles techniques développées par les faussaires. C'est pourquoi nous accueillons favorablement l'initiative de Bernard Fialaire. La création d'un registre des faux faciliterait le travail des enquêteurs. la proposition de loi alourdit considérablement les peines et prévoit des circonstances aggravantes lorsque les faux sont réalisés au détriment d'une personne publique ou commis en bande organisée. La rédaction proposée élargit enfin la qualification du faux. Nous serons toutefois très attachés à trouver un meilleur équilibre entre la protection des droits patrimoniaux des collectionneurs et des marchands d'art et la protection des artistes. Le droit d'auteur est un corollaire de la liberté d'expression artistique. Il ne doit pas devenir une entrave à la création. C'est pourquoi nous présenterons des amendements destinés à exclure la destruction des oeuvres jugées comme faux, en considérant que ces dernières peuvent disposer d'une valeur intrinsèque, autonome de l'identité de l'artiste, même faussaire. D'autres pistes pourraient être envisagées, comme la mise sous séquestre automatique. De la même manière, nous souhaitons préserver la capacité des artistes à créer leur nom d'emprunt et leur permettre de garder secrètes leurs techniques de fabrication. La protection des artistes doit être replacée au centre de nos préoccupations de législateur, alors que le marché, toujours plus fort, s'est encore renforcé pendant la crise sanitaire. Entre 2007 et 2013, 30 % des expositions personnelles proposées par les grands musées américains ont ainsi été consacrées à des artistes représentés par seulement Certains artistes se battent contre cette tendance. Je pense à Banksy, dont l'une des oeuvres a été détruite en pleine salle des ventes. Je pense aussi, avant lui, à Marcel Duchamp présentant un urinoir comme une fontaine ou à René Magritte qui nous interpellait avec son célèbre tableau, accompagné de la

De leur capacité à nous illusionner dépend notre capacité à nous émerveiller. À nous de veiller à ce que leur liberté d'expression demeure entière. La parole

La technologie a complètement transformé le marché et les moyens par lesquels les oeuvres d'art sont créées et vendues. On a vu l'apparition et l'essor de nouvelles technologies telles que la 3D ou les NFT, ces jetons numériques qui ont permis de numéroter et de rendre chaque oeuvre unique. Malheureusement, la loi Bardoux et le droit commun en général ne se sont pas toujours enrichis ni adaptés à ces changements. De fait, les artistes sont de plus en plus exposés aux fraudes et à la contrefaçon. Ainsi, ceux qui vendent leurs oeuvres en ligne sont très vulnérables aux escroqueries et aux pirates informatiques, tandis que ceux qui vendent leurs oeuvres dans des galeries peuvent être sujets aux pratiques douteuses de certains professionnels. Aujourd'hui, la loi Bardoux n'offre aucune protection aux artistes contre le vol de leurs oeuvres. C'est particulièrement préoccupant, à l'heure d'internet et des réseaux sociaux. Ils sont donc souvent contraints de recourir à des moyens légaux coûteux pour se défendre contre ces pratiques. Cela pousse parfois certains d'entre eux à exercer une surveillance constante. Or les auteurs et leurs ayants droit n'ont pas toujours les moyens matériels, humains et financiers pour lutter seuls face à ce phénomène en constante expansion. Personne ne remet en cause la nécessité d'actualiser la loi ni de compléter notre arsenal législatif en la matière. Il faut mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle, mieux protéger les artistes contre les pratiques abusives, leur permettre de mener leurs activités avec plus de sécurité et de confiance et encourager évidemment une plus grande transparence dans le marché de l'art. Cette proposition de loi apporte des réponses utiles pour lutter contre les fraudes causant des préjudices aux artistes et aux acquéreurs d'oeuvres d'art. Elle définit une nouvelle infraction pénale et procède à une refonte de la répression,

d'une part, les fraudes portant directement sur l'oeuvre d'art- la réaliser ou la modifier -, d'autre part, les fraudes réalisées autour de l'oeuvre d'art- la présenter, la diffuser ou la transmettre à titre gratuit ou onéreux.

Sur le volet répressif, les peines étaient jusqu'alors insuffisantes. L'établissement de circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis par des professionnels du marché de l'art et lorsque le préjudice est subi par une institution patrimoniale publique était indispensable. En parallèle, l'enjeu est d'éviter la remise sur le marché de l'oeuvre falsifiée, tout en veillant à l'équilibre avec le risque de destruction d'une oeuvre sur laquelle il y aurait toujours un doute. Ainsi, la création d'un registre de fraude artistique contribuera à cette lutte. Nous ne doutons pas que les résultats des travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique enrichiront ce texte au cours des prochaines étapes de la navette parlementaire. Le travail mené en commission sous votre houlette et non votre baguette, monsieur le rapporteur, a permis de préciser et de clarifier le texte initial, le rendant ainsi plus opérationnel. Comme l'a dit Max Brisson, le groupe Les Républicains votera la loi Fialaire. Pardon pour le plagiat

recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes ». La réécriture proposée dans cet amendement est beaucoup plus large que ce que prévoit le droit actuel. Elle vise non seulement la vente, mais également la présentation, la diffusion ou la transmission à titre onéreux d'oeuvres ou L'interdiction faite de tromper par quelque moyen que ce soit sur l'identité du créateur ne doit pas être prise à la légère, car elle pourrait se retourner contre les artistes qui se décideraient à créer sous un nom d'emprunt. Ce fut par exemple le cas de Marcel Duchamp, quand il signa sa fontaine « R. Mutt », de Romain Gary, dissimulé derrière Émile Ajar, ou encore des Daft Punk, dont on ne connaît pas- du moins, c'est mon cas -la véritable identité. Il faut absolument protéger ce droit. C'est pourquoi nous proposons une réécriture de cet article afin d'exclure totalement ce risque et de clarifier une zone d'ombre rédactionnelle. Quel est l'avis de la commission ? Madame de Marco,

Néanmoins, votre amendement tend à supprimer toute référence à la notion de tromperie, qui figurait dans le texte adopté par la commission. Or cette notion me paraît essentielle à la définition de l'infraction pénale, l'on veut garantir la répression des seules manoeuvres frauduleuses et éviter justement de brider la liberté de la création. La rédaction de votre amendement celui d'interdire certaines pratiques artistiques, à commencer par la copie, dans la mesure où la simple intention d'attribuer l'oeuvre à un autre pourrait être sanctionnée. J'ajoute que la rédaction du texte de la commission ne remet pas en cause, à mes yeux, la possibilité, pour un artiste, d'utiliser un pseudonyme. On pourrait d'ailleurs considérer que les différents pseudonymes utilisés par un artiste sont partie intégrante de son identité d'artiste. L'infraction doit permettre de sanctionner les seuls cas dans lesquels l'identité d'un créateur, qu'il s'agisse de son vrai nom ou de son pseudonyme, a été usurpée.

amende et à de la prison tout artiste qui présenterait, diffuserait ou transmettrait une oeuvre en trompant sur sa composition. Je comprends l'intention de protéger les collectionneurs de mobilier de collection par exemple, mais cette écriture me paraît trop large et susceptible de porter atteinte à la liberté artistique qui justifie parfois de faire passer un matériau pour un autre ou de cacher la nature des matériaux. Selon moi, ce n'est pas la matière utilisée qui fait l'oeuvre, mais c'est l'agencement recherché par l'artiste, sa technique. On attribue souvent à Picasso cette citation : « Certains peintres transforment le soleil en un point jaune. D'autres transforment un point jaune en soleil. » Laissons donc les artistes nous illusionner avec la matière qui leur plaira.

Je souhaite vous rassurer sur le fait que l'objectif n'est nullement de contraindre les artistes à dévoiler leurs secrets de fabrication artistique, lorsqu'ils mettent en vente leurs oeuvres. En mentionnant les tromperies sur la composition, c'est bien, par exemple, les tromperies sur les matières utilisées que nous avions en tête, si celles-ci sont mentionnées, ou encore les restaurations ou reconstitutions excessives qui ont pour effet de faire perdre à une oeuvre ou à un objet d'art son caractère authentique. aussi penser à la fabrication de faux meubles, en utilisant des matériaux anciens. Il me semblerait regrettable que des escroqueries de ce type ne puissent pas être sanctionnées. D'ailleurs, le terme de « composition » est repris du décret Marcus qui impose aux vendeurs la délivrance de certificats d'authenticité contenant les « spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue

Elle prévoit en effet de permettre au juge d'ordonner la destruction d'un bien culturel saisi sur le fondement du nouvel article L. 112-28 du code du patrimoine. Une telle disposition est déjà prévue par le code pénal pour les biens dangereux ou nuisibles et le Conseil constitutionnel a rigoureusement encadré cette faculté donnée au juge dans le cas des armes à feu. Il me paraît donc disproportionné de l'étendre aux biens culturels, même frauduleux. Je comprends l'intention du rapporteur, mais je pense que des solutions alternatives devraient être recherchées, comme l'automaticité de la mise sous séquestre ou des techniques de marquage des châssis d'époque utilisés par les faussaires. Nous nous sommes entretenus avec les représentants de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), qui ont reconnu que des solutions moins abruptes pourraient être envisagées.

commission ? Madame de Marco, vous vous inquiétez de la possibilité offerte au juge par la proposition de loi de prononcer la destruction de l'oeuvre

Il ne serait pas acceptable qu'une oeuvre d'art simplement revêtue d'une signature apocryphe soit détruite, car, à l'exception de cette signature trompeuse, elle reste l'oeuvre originale d'un artiste qui mérite d'être rétabli dans ses droits. Surtout, si la signature peut être retirée, il n'y a aucune raison que l'oeuvre ne puisse pas être remise sur le marché. C'est la raison pour laquelle le texte de la commission se contente de donner un un panel d'outils au juge pour permettre de retirer l'oeuvre d'art litigieuse du marché, mais celui-ci ne sera en aucun cas contraint d'en faire usage : il conservera sa liberté d'appréciation en fonction des circonstances. J'ajoute

Le code général de la propriété des personnes publiques autorise déjà la destruction des oeuvres falsifiées déclarées comme telles en application de la loi Bardoux. Il n'y a donc pas vraiment de changement par rapport au droit existant, si ce n'est qu'aujourd'hui cette décision appartient entièrement à l'administration des domaines,

que le faux. En matière d'art, c'est particulièrement exact et tout le mérite de ce texte, notamment dans son article 1, est d'arriver à définir à partir de quel moment une intention devient malveillante et un acte répréhensible.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Merci

de construction de logements et de réindustrialisation de la France. Pour répondre à une partie du problème, il est proposé, pour certains projets dont l'intérêt est majeur- réindustrialisation, logement social, etc. -, de disposer d'un recours auprès de l'autorité compétente de l'État pour obtenir leur sortie de l'enveloppe d'artificialisation, lorsque leur comptabilisation serait de nature à compromettre de manière irréversible l'atteinte des objectifs généraux. Dans cette hypothèse et pour éviter toute péréquation inéquitable sur les territoires voisins, leur emprise serait sortie de la trajectoire ZAN nationale et régionale et soldée dans le cadre du bilan périodique du ZAN par tranche de dix ans jusqu'à 2050.

et à l'élargir à l'ensemble des projets concourant à la production et au stockage d'énergies renouvelables. Après la date de 2031, les collectivités seront dans une impasse. En effet, le développement des énergies renouvelables dans leur territoire, sur leur initiative ou non, pourrait grever leur capacité d'artificialiser leurs sols. Il s'agit donc d'exclure ces réalisations du calcul des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation, afin de ne pas entraver la capacité de nos collectivités à développer ces projets, tout en permettant d'autres réalisations, pour les activités économiques ou pour l'habitat. Quel est l'avis de la commission spéciale ? Je comprends

compétents en matière d'urbanisme, entraînant ainsi une délibération motivée du conseil régional pour refuser ou accepter chacune des demandes, après avis de la conférence régionale de la gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. Cette procédure, lourde et contraignante, place les régions dans une situation de justification permanente. Elle crée aussi de l'instabilité, en raison de la possible modulation- sans fin et à la hausse -de l'enveloppe régionale, ce qui est incompatible, comme vous le savez, avec l'atteinte de l'objectif de 50 %, fixé à l'échelle régionale. C'est pourquoi le sénateur M. Étienne Blanc souhaite supprimer cet article.

Les communes et les EPCI dotés de la compétence urbanisme seront donc force de proposition dans l'identification de ces projets. Il est également prévu par cet article que la région se prononce par délibération motivée en conseil régional sur les suites à donner à ces demandes.

cet amendement vise à supprimer la délibération motivée du conseil régional prévue pour chaque projet, afin de ne pas alourdir les débats et afin que

M. Jean-François Longeot. Cet amendement, déposé par Michel Canévet, vise à permettre la prise en compte des projets d'intérêt supracommunal dans la fixation des objectifs de réduction de l'artificialisation, à l'échelle d'un EPCI.